Non c'est pas de. L'ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2022. Et la parole est à madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargé de l'Europe. M.. La ministre, c'est à vous.-- Madame la présidente, monsieur le président de la commission des Affaires étrangères. De la Défense et des forces armées. Monsieur le président de la commission des Affaires européennes. Monsieur le président de la commission des finances. Mesdames, et messieurs les sénateurs.-- Fidèle à nos traditions. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver afin de vous présenter. Et d'échanger. Comme de coutume avant chaque conseil européen. Sur les principaux sujets qui seront traités. La guerre en Ukraine continuera bien sûr d'être le sujet le plus brûlant. Mais je pense aussi naturellement à la crise énergétique et à la situation économique ces 2 dernières étant comme vous le savez intrinsèquement liées.-- Ce constat est partagé par tous. J'ai eu l'occasion de le dire sur vos bancs lors de l'examen du prélèvement sur recettes le 17 novembre dernier. Je crois aussi que votre commission a pu entendre le même jour une communication du sénateur Patrice Joly portant sur le cadre financier pluriannuel au défi de la guerre en Ukraine.-- Le Conseil européen sera également marquée par des discussions d'une part sur la sécurité et la défense. Et d'autre part sur notre politique étrangère. Il y a aussi des échanges prévus sur les relations avec le voisinage sud. Les États-Unis et les Balkans occidentaux. Enfin, il sera précédé d'un sommet entre l'Union européenne et l'Asean.-- Comme vous le savez, la situation évolue tous les jours et les positions que je vais vous exposer sont bien sûr encore susceptible d'évoluer à l'aune des événements que vous connaissez et des concertations qui sont conduites entre Europe en ce qui concerne la guerre en Ukraine qui continue avec les poursuites, ces dernières semaines d'une stratégie de frappe brutale de la Russie contre les infrastructures civiles énergétiques ukrainiennes.-- Affaiblir l'Ukraine par un froid par le enfin dans la fin, c'est la stratégie de Vladimir Poutine. Il faut donc maintenir notre soutien à l'Ukraine dans toutes ses dimensions et à long terme l'urgence étant évidemment aujourd'hui de permettre aux Ukrainiens de passer l'hiver.-- C'est pour cela que le président de la République a décidé, avec le président ukrainien Zelensky d'organiser une conférence sur la résilience de l'Ukraine, le 13 décembre à Paris. Afin de répondre aux besoins de court terme dans le domaine de la résilience des infrastructures civiles.-- Également afin de structurer notre aide financière à l'Ukraine à long terme, la Commission a proposé la mise en place d'un soutien financier sous forme de près. De 18 milliards d'euros pour l'Ukraine pour l'année 2023. Aujourd'hui, il n'a pas été possible de parvenir à un accord au Conseil des ministres de l'Économie et des Finances, mais nous sommes confiants sur notre capacité à y parvenir avant la fin de l'année. Afin que les premiers versements puissent avoir lieu dès le mois de janvier.-- Il en va de la crédibilité, l'Union européenne et des engagements pris par nos chefs d'État et de gouvernement. La situation énergétique maintenant comme vous le savez, reste préoccupante. je salue une nouvelle fois les travaux de votre commission. Monsieur le Président rap. Et notamment l'organisation de la table ronde de haute tenue le 16 novembre dernier sur les ambitions européennes et les chocs économiques actuelles.-- Nous devons nous appuyer sur tous les règlements adoptés pour accélérer la réduction de notre dépendance à l'égard de la Russie et des énergies fossiles.-- Évidemment nous saluons les efforts de la commission, elle a fait trois nouvelles propositions législatives susceptibles de répondre à une partie des enjeux liés à notre sécurité énergétique.-- Ces propositions permettraient d'agir partiellement sur le prix du gaz, de mettre en place une plateforme conjointe de gars d'achat conjoint pardon de gaz et de renforcer notre solidarité énergétique.-- Nous nous félicitons aussi qu'un accord politique était trouvé lors du Conseil Énergie extraordinaire du 24 novembre. Sur les 2 règlements, présenté le 18 octobre et le 9 novembre. Même si leur adoption formelle n'interviendra que la semaine prochaine.-- Je crois qu'il faut quand même le dire, l'ensemble de ces mesures ne répond toutefois pas à l'urgence de la situation en dépit de la nouvelle proposition du 22 novembre portant sur un marché correctif mécanismes correctifs sur le marché du gaz.-- Ce texte prévoit certes une forme de plafonnement sur une partie des prix du gaz mais dans des conditions qui nous semble excessivement restrictives. Il doit donc encore gagner en crédibilité et en pertinence dans la situation actuelle. Il est essentiel vraiment essentiel que nous envoyons un signal fort au marché.-- Et puis nous devons aller plus loin pour faire baisser les prix du gaz et de l'électricité, le président l'a d'ailleurs demandé au dernier conseil européen.-- nous allons continuer d'appuyer des mesures qui permettent de faire baisser les prix à court et moyen terme, avec une réforme du marché de l'électricité.-- Il est également impératif que nous apportions des réponses budgétaires coordonnées afin de lutter contre l'inflation tout en préservant la croissance.-- Nous attendons des propositions de la Commission européenne pour avancer sur la mise en oeuvre de mécanisme européen de solidarité financière. Afin d'éviter toute fragmentation économique entre les États de l'Union. Le Conseil européen abordera ensuite les enjeux de sécurité et de défense. Le renforcement de l'industrie de défense européenne figure parmi les priorités du Conseil européen et ce dans la continuité des engagements qui ont été pris lors du sommet de Versailles.-- La Commission européenne a annoncé lundi avoir débloqué un 1er financement de 1,2 milliards d'euros du Fonds européen de la défense pour la prochaine génération d'avions de combat des projets de char et de navires et le développement de technologies militaires.-- C'est ainsi, 61 projets qui vont être cofinancée pour fournir des capacités de pointe à nos forces armées par ce fonds européen de défense qui est dotée comme vous le savez de 7 9 milliards d'euros pour la période 2021 2027.-- Là aussi il nous faut aller plus loin. Il est nécessaire d'avancer rapidement sur le règlement qui crée un instrument d'urgence pour faciliter l'acquisition conjointe de matériel militaire les dire pas. Il est en cours de négociation. Puis sur la construction d'un instrument pérenne les. Ces instruments vont être déterminants pour nous aider à structurer la demande et donc à donner davantage de visibilité à nos industriels.-- Il doit aussi être conçu d'une manière qui nous aident à réduire nos dépendances sur des technologies et des chaînes d'approvisionnement contrôlés par des États non-européens.-- La résilience et la cybersécurité des entités critiques européenne dans la lignée seront aussi à l'ordre du jour.-- La palette de d'instruments que nous sommes en train d'adopter à cet égard constituera un pilier de notre stratégie numérique est également l'une des clés d'une souveraineté affirmé.-- Une mise en oeuvre rapide et efficace sera évidemment importante. Pour avoir une pour la notre résistance Fax aux actes malveillants à l'encontre de nos infrastructures critiques. bien sûr ces objectifs ne doivent pas occulter le besoin de renforcer la coopération avec nos partenaires internationaux, en particulier les plus exposés.-- Cette coopération je crois plus que jamais, elle doit être un levier important de notre stratégie en matière de cybersécurité et de résilience.-- Enfin ce conseil européen sera l'occasion d'un soutenait d'assurer la soutenabilité de la Facilité européenne de paix.-- Comme vous savez, elle a été mobilisés de manière massive inattendu pour soutenir l'Ukraine.-- Et l'Union européenne a su utiliser à des fins nouvelle un instrument qui avait été initialement conçu pour la gestion de crise et l'accompagnement des missions de formation.-- Évidemment nous ne pouvons que nous féliciter de cette capacité d'adaptation de l'Union européenne puisqu'aujourd'hui c'est grâce à la FEPS que l'UE que l'Union européenne est devenu un acteur majeur sur le plan militaire dans le conflit ukrainien. Avec 3 milliards d'euros mobilisé à ce titre.-- Toutefois cela fait peser un risque sur la soutenabilité de l'instrument et notamment sa capacité à continuer de porter l'ambition initiale de l'instrument.-- C'est pourquoi le Conseil européen sera l'occasion d'acter un réabonnement de l'instrument d'une manière qui suivent au plus juste ses besoins réels.-- Comme je vous disais en introduction, le Conseil européen se penchera aussi sur nos relations avec le voisinage sud, notamment en préparation d'un sommet prévu pendant la présidence espagnole du Conseil au 2ème semestre 2023.-- Ces discussions sont extrêmement importantes et nous avons eu l'occasion d'en d'en débattre ici. Dans le contexte de l'agression russe en Ukraine, il est. Essentiel de lutter contre le narratif russe dans la région. Et de poursuivre notre soutien à la prospérité et à la stabilité de cette région dont les soubresauts nous affecte directement.-- À Barcelone, le 24 novembre dernier, les ministres de l'Union européenne et des pays du voisinage sud. pour moi, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte, Jordanie, Liban, Israël et Palestine. Ont échangé sur les pistes de coopération pour répondre au double défi posé par l'agression russe en Ukraine.-- Celui de la sécurité alimentaire qui est mise en péril dans plusieurs pays du voisinage sud en particulier en Tunisie, au Liban et en Égypte et qui requiert la poursuite de notre action. À leurs côtés. Et aussi celui de l'énergie à l'heure où cette guerre vient renforcer l'intérêt de diversifier nos approvisionnements et d'inscrire nos partenariats avec les pays du sud, dans la durée.-- L'inscription du point voisinage sud à l'agenda et du Conseil européen contribuera donc à ses objectifs en maintenant la dynamique de l'Union européenne en faveur d'une politique méditerranéenne ambitieuse et positive.-- S'agissant des relations extérieures. Le Conseil européen va être précédé par un sommet entre l'Union européenne et l'Asean le premier. Au niveau des chefs d'État et de gouvernement des 2 blocs. Il s'agit d'un moment essentiel pour poursuivent l'engagement européen renforcé dans l'Indopacifique et mettre en oeuvre le partenariat stratégique UE-Asean qui, comme vous le savez a été signé en 2020, notamment dans le cadre de projets financier avec l'initiative européenne globaux Le Conseil européen devrait enfin revenir sur 2 aspects d'actualité. D'une part nos relations avec les États-Unis dans un contexte qui est marqué par l'adoption de ligne flèche réduction Act. Et d'autre part les relations de l'Union avec les Balkans occidentaux dans un contexte marqué par la demande du statut de candidat de la Bosnie. Sur les relations avec les États-Unis. Ensuite le Conseil européen il viendra en discuter après une séquence qui comme vous l'avez vu a été chargé. Le président de la République s'étant rendus aux États-Unis du 29 novembre au 3 décembre pour cette 2ème visite d'État à Washington la première visite d'État de l'administration Biden, ce qui est le signe de la densité de notre relation bilatérale.-- Il a porté un message très clair. En étroite relation avec nos partenaires européens. Sur les gens je énergétique et sur les enjeux commerciaux.-- La 3ème réunion du Conseil, commerce et technologie UE-États-Unis qui s'est déroulée hier et avant-hier a aussi permis à l'Union européenne d'approfondir ses messages. Comme vous le savez, c'était ça enceinte est importante pour aborder en partenaires les défis communs auxquels nous faisons face.-- Et puis concernant le projet d'une flèche une réduction Act l'intention en matière climatique des États-Unis est évidemment louable. Il faut s'en féliciter, mais les modalités prévues par ce dispositif comme vous le savez, vont créer des distorsions de concurrence pour nos entreprises et notre activité.-- les mesures prises dans ce cadre sont absolument contraires à l'esprit de coopération transatlantique. Nous devons identifier des solutions qui préserve pleinement les intérêts européens et c'est ce qu'a dit très clairement, le président de la république et ce sont les les messages qui ont été passés lors du CCT. La task force qui a été mis en place au niveau de la Commission doit nous permettent de trouver rapidement une solution négociée conforme aux intérêts européens et vous pouvez compter sur nous pour être très attentif à ces résultats.-- Cependant. Il nous semble que l'Union européenne doit se préparer dès à présent à l'éventualité d'une absence de prise en compte des demandes européennes ou ne dure une reprise vraiment a minima de celle-ci. Et l'Union européenne doit se préparer pour être en mesure d'agir et d'envoyer des signaux efficace aux entreprises avant la fin de l'année.-- Il faut notamment avancé très vite sur la proposition faite paru sur la Dans son discours sur l'état de l'union de création d'un fonds de souveraineté européen et je crois que nous devons également étudier comment les instruments anti-subventions mises en place pendant la présidence française de l'Union européenne peuvent trouver à s'appliquer.-- Enfin le Conseil européen traitera de la question des Balkans occidentaux.-- Comme vous savez, la France est résolument en faveur du processus d'adhésion des Balkans occidentaux à l'Union européenne et nous n'avons pas compté nos efforts en ce sens pendant la présidence pendant notre présidence du conseil, comme en témoigne notamment notre engagement en faveur de la résolution du différend bulgaro-macédonien. Qui a permis la tenue des premières conférence intergouvernementale d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. En juillet dernier.-- J'ai d'ailleurs eu l'occasion de me rende récemment en Albanie mais Macédoine du Nord pour confirmer aux gouvernements de ces pays notre implication dans la durée. Pour poursuivre cet élan. L'organisation du sommet Union européenne Balkans occidentaux de Tirana aujourd'hui même est une excellente opportunité, en particulier pour marquer notre solidarité et notre soutien dans le contexte actuel.-- L'Union européenne et d'des d'ores et déjà pleinement engagée aux côtés des Balkans occidentaux et ce sommet a été l'occasion de montrer concrètement nos actions dans la région qui doivent être poursuivis et amplifiés afin que les pays des Balkans occidentaux retire des bénéfices concrets des efforts qu'ils auront consentis. On peut penser par exemple au paquet de soutien énergétique d'un milliard d'euros à la poursuite de la mise en oeuvre du plan économique et d'investissement à des initiatives dans le domaine cyber qui ont déjà vu le jour. Au projet de réduction progressive des frais d'itinérance téléphonique entre l'Union européenne et des Balkans occidentaux discuter aujourd'hui même. En Bosnie-Herzégovine, nous espérons la formation rapide des gouvernements à tous les niveaux, à la suite des dernières élections, elles étaient le 2 octobre. Vous vous en souvenez. Il s'agit bien évidemment d'une étape indispensable pour la fonctionnalité des institutions et la poursuite des réformes.-- Quant à la question de l'octroi du statut de pays candidat. Le Conseil européen prendra une décision la semaine prochaine en prenant en compte tous les paramètres en jeu, que ce soit le contexte géopolitique, mais aussi les progrès du pays dans la mise en oeuvre des réformes.-- La poursuite du chemin européen d'Apps Hosni Herzégovine dépend avant tout de la volonté politique des dirigeants bosniens et ceux-ci doivent commencer dès à présent à mettre en oeuvre les réformes identifiées par la commission.-- Vous le voyez j'espère vous en avoir convaincu messieurs les prix. Madame la présidente, messieurs les présidents, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. C'est un programme chargé pour ce Conseil européen. Il témoigne de l'énergie de l'Union européenne pour faire face ensemble aux conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine mais sans laisser de côté l'ensemble des sujets de long terme qui font notre unité, je vous remercie. Merci madame la ministre, hein. La parole est à monsieur Pascal Alizart vice-président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour cinq minutes.-- Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Conseil européen qui se tiendra le 15 décembre prochain, ce sera le 1er depuis la libération de Kherson par les troupes Le succès de la contre-offensive lancée par l'État-Major ukrainien en septembre ne saurait masquer les nombreuses incertitudes qui continuent d'obscurcir le Champ de bataille, la guerre déclenchée en février dernier par l'agression russe sur le territoire ukrainien dure depuis plus de 9 mois. D'ores et déjà, cette guerre est inédite par son ampleur, son intensité sur notre continent depuis la fin de la guerre froide. Il existe malheureusement un risque réel pour qu'elle s'installe dans la durée. S'il est difficile de prédire ce que sera l'avenir de cette guerre du constatons déjà sur le théâtre d'opération l'importance de la mobilisation des Européens en faveur de la liberté du peuple ukrainien. Au lendemain du 24 février notre Union européenne a fait la preuve de sa capacité à s'unir et à se mobiliser y compris sur la scène géopolitique internationale depuis cette date, le total des livraisons des livraisons d'armes létales et non létale. Assurée par les États membres au bénéfice des soldats ukrainiens dépasse les 8 milliards d'euros. Cette somme n'atteint certes pas les 19 milliards de dollars de l'aide américaine mais elle représente une contribution substantielle et surtout décisive à l'effort de guerre de l'Ukraine. Les soldats ukrainiens font chaque jour la démonstration de l'importance intact des forces morales pour prendre la supériorité sur le terrain. Il est de notre devoir de continuer de leur apporter un soutien financier et capacitaire à la hauteur de leur résistance héroïque. Pour ce faire nous devons à tout prix préserver l'unité qui caractérise l'Union européenne depuis le début de la guerre. Or, à l'échelle de l'Union les instruments que nous avions imaginé pour une période de paix ne sont plus adaptées pour cette période de guerre la Facilité européenne pour la paix a démontré depuis sa création 2021 sa pertinence et sa souplesse d'utilisation. Mais le montant de 5,7 milliards d'euros que nous avions initialement prévu se révèle largement en deçà des besoins. La situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons exige d'y apporter des réponses exceptionnelles le versement des aides prévues par la sixième enveloppe avalisé lors du sommet de Prague en octobre portera à plus de 3 milliards le financement de l'aide aux armées ukrainiennes portées par cette Facilité européenne pour la paix le refinancement de cet instrument financier devient donc une urgence. Le retour de la guerre sur notre continent justifie pleinement la mobilisation de crédits exceptionnels pour cette opération. Nous devons nous mobiliser pour que l'Union continue de s'appuyer sur un instrument suffisamment solide pour financer l'aide militaire décidée en commun. Au-delà de cet enjeu de court terme sur lesquels les chefs d'État et de gouvernement devront trouver rapidement un compromis praticable la coopération européenne de défense doit répondre à des enjeux de long terme la boussole stratégique européenne bien évidemment la mobilisation des gouvernements au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine s'est traduite par une hausse générale des Budgets de défense au sein de l'Union. Mais si nous n'y prenons pas garde cette hausse pourrait avoir des effets. De renforcer l'empreinte des industries d'armement américaines en Europe, l'ambition française d'une d'une autonomie stratégique européenne ne sauraient se satisfaire d'un tel résultat. Ce que nous devons promouvoir dans le sillage de la boussole c'est un renforcement de nos dépenses en commun que cela soit pour financer de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la défense ou pour financer des achats d'équipement, les statistiques les plus récentes sont inquiétantes dans ce domaine et font état d'une proportion des acquisitions communes de matériel militaire qui atteint seulement 18% en 2021, c'est 2 fois moins que l'objectif fixé dans le cadre de la boussole stratégique de 35% des équipements en commun. Dans ce contexte, la défense collective de l'Europe ne pourra être assurée qu'à la condition de répondre aux défis soulevés à court terme et à moyen terme par le retour de la guerre sur notre continent. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous serons attentifs à ce que la France soutienne les solutions qui permettront à l'Europe de se doter de l'autonomie stratégique que les circonstances exigent. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Albéric de Montgolfier 1000 vice-président de la commission des finances pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. Il est difficile d'évoquer le Conseil européen qui se tiendra d'ici 10 jours sans prendre en compte le Conseil Affaires économiques et financières qui s'est tenu ce matin même. Vous serez donc pas étonné Madame la Ministre que ma première question porte sur les résultats de cette réunion. Pouvez-vous nous ont précisé les conclusions, je pense en particulier l'avancement à l'état d'avancement du dossier des ressources nouvelles auxquelles auxquelles la commission des finances est très attentive puisqu'il conditionne les modalités de remboursement du plan européen.-- Plus précisément, il semble que le mécanisme d'abus justement carbone aux frontières fasse encore l'objet de divergences alors qu'il doit entrer en vigueur dès 2023. Un mois que vous nous annonciez à un report de cette échéance. Peut-être ce soir. Qu'en est-il du Champ d'application du mécanisme. Qu'en est-il de la suppression des quotas gratuits. Pouvez-vous également nous indiquer si l'utilisation des revenus issus de ce mécanisme est désormais stabilisée en clair nous dire c'est cas le niveau de ressources viendra abonder le budget européen. La réforme du marché du carbone me fournit une transition pour aborder un point de l'ordre du jour du prochain conseil européen qui préoccupe tout particulièrement. La commission des finances, c'est-à-dire les liens entre la crise énergétique et notre économie.-- Cela a déjà été souligné mais j'y insiste, l'évolution du cours du gaz inédite depuis le début de l'année 2021. Après tout à fait considérable dans son ampleur et dans l'histoire européenne. Cette hausse se répercute évidemment sur les consommateurs sur les entreprises. C'est la raison pour laquelle la commission des finances, avait proposé l'adoption sans modification de l'article 12 quater du projet de loi de finances pour 2023, adopté cet après-midi qui vise à prolonger les dispositifs de bouclier tarifaire pour le prix de le gaz et les prix de l'électricité, l'année prochaine. Sans un prolongement de ce mécanisme. Les prix de l'est connu de l'énergie aurait connu une évolution insupportable pour les acteurs économiques, il ne peut évidemment être évaluée sans prendre en compte les contextes économiques et le contexte européen, ce qui me conduit à vous poser 3 questions. Première question, quelles sont les perspectives d'accord sur le plafonnement du prix du gaz. Qu'en est-il de la réforme à venir du marché de l'électricité et quel sera l'impact du plafonnement du prix du pétrole russe plafonnement qui a été décidé, comme vous le savez, la fin de la semaine dernière, conjointement avec les pays du G7 et avec l'Australie.-- La crise unique énergétique me conduit à aborder également une préoccupation majeure pour les mois à venir puisque depuis 30 ans, nous vivons dans l'idée que l'inflation avait pratiquement disparu, mais nous le savons 2022 a bouleversé cette croyance et l'inflation dépasse aujourd'il 10% en moyenne dans l'Union européenne. Sur le plan financier, on peut évidemment s'interroger sur l'impact de ce choc exogène sur la mise en oeuvre de la facilité pour la reprise et la résilience en effet. Les montants disponibles avait été fixé début 2021 puis ajuster au 30 juin dernier mais aujourd'hui ne sont-ils pas dépasser, dans la mesure où la hausse des prix fous je touche très fortement tous les États européens. Il n'est pas je disais en moyenne 10% mais dans certains états, comme les pays baltes, c'est 20% d'inflation. À l'inverse, ne croyez-vous pas que dans ce contexte de dégradation de la situation économique et financière. Certains États éprouvent des difficultés à honorer leurs engagements quant au financement du budget européen. Si la hausse des prix. Des conséquences une instamment une conséquence mécanique immédiate, celle d'accroître les recettes de TVA. Les perspectives de récession ne peuvent qu'avoir qu'un impact négatif tant sur le montant reçu qu'au titre, notamment au titre des droits de douane. Vous savez que leurs droits de douane sont la ressource propre traditionnelles d'union que sur le revenu national brut qui représente la principale source de financement du budget européen. Ce contexte général, en clair va-t-il se traduire par une accélération de la mise en chantier de la révision du cadre financier pluriannuel 2021 2022. Tels étaient les quelques questions Madame la Ministre que je souhaitais vous posez au nom de la commission des finances, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-François Rapin, président de la commission des Affaires européennes pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la Ministre, mes, mes chers collègues. Donc, Conseil. Européen le 15 décembre Madame la Ministre donc une journée destinée finalement à à plusieurs. Plusieurs Les 3 sujets qu'on peut évoquer. Seront des sujets directement liés. À la crise en Ukraine. L'énergie des relations transatlantiques et un point particulier sur. La guerre et ses conséquences.-- Comme depuis plus de neuf mois cette prochaine réunion sera dominée malheureusement par la guerre en Ukraine où la Russie accentue la pression sur les civils en violation enfin flagrante des règles sont dans l'ordre international. Nous comptons bien entendu sur le Conseil européen pour renouveler le soutien de l'Union à l'Ukraine sur tous les plans et vous l'avez précisé Madame la Ministre tout à l'heure, surtout au plan financier bien sûr mais diplomatique et militaire c'est évident comme humanitaire, nous y reviendrons. Et pour obtenir que la Russie assume la responsabilité pleine et entière des crimes qu'commet à ce sujet. Nous venons de recevoir au Sénat une délégation de parlementaires ukrainiens menés par Maria. CEVA, venu à Paris pour plaider en faveur de la mise en place d'un tribunal spécial chargé de juger le crime d'agression constitué par l'invasion russe. Il est très important d'évaluer les différentes solutions juridiques envisageables pour que justice soit rendue dans les meilleures conditions d'impartialité et de sécurité juridique sans quoi et on le sait aucune paix durable ne pourra jamais se construire en Ukraine. Dans ce contexte, le soutien public récemment apporté par la présidente de la Commission européenne à l'hypothèse du tribunal spécial réclamée par l'Ukraine ne peut manquer d'interroger Madame la Ministre le Conseil européen ne serait-il pas plus légitime pour s'engager au nom de l'Union sur cette question juridiquement complexe et politiquement sensible. Le 2ème point. La crise énergétique. Ce sera le 2ème sujet qui en lien avec le Premier s'imposera au Conseil européen, lors de sa prochaine réunion. L'objectif à court terme est double, à la fois cesser d'alimenter la Russie par nos achats d'énergie et amortir le choc économique et sociale que provoque la hausse des prix de l'électricité et plus globalement l'inflation. Le sujet reste préoccupant malgré l'accalmie apparente que l'on doit aux températures clémentes à l'approvisionnement soutenu en GNL et à la quasi saturation des capacités de stockage européenne sur le long terme. L'Europe a besoin d'une énergie abondante, bon marché et décarboner la commission des Affaires européennes travaillent avec celle des affaires économiques sur les réformes envisageables du marché de l'électricité européen pour y parvenir. À cet égard l'impulsion donnée par le Conseil européen des 20 et 21 octobre dernier reste inaboutie. Même s'ils s'accordent pour réduire la consommation d'électricité. Taxer les superprofits. Les États restent divisés sur les décisions structurantes que la crise exige de prendre et il continue d'avancer en ordre dispersé avec le risque d'effets pervers et de distorsion de concurrence importante entre. Nos industries ne peuvent pâtir plus longtemps des initiatives prises par d'autres États membres qu'il s'agisse du mécanisme ibérique ou des aides d'État dont bénéficient leurs concurrentes allemandes dans quelle mesure le mécanisme temporaire de correction des prix du gaz que propose la Commission européenne peut-il sauver la compétitivité de nos entreprises. Vous l'avez évoqué tout à l'heure mais je pense que. Ça nécessite des réponses plus précises encore. C'est le même souci qui m'amène à évoquer un sujet que vous avez partagé avec nous l'inflation réduction Act cet arsenal législatif très puissants, dont les États-Unis se sont dotés pour pour stimuler leur économie au prétexte de la transition verte lors de sa récente visite aux États-Unis, le président de la République n'a pu que déplorer le déséquilibre concurrentiel qui en résultent pour notre côté de l'Atlantique. Il est urgent que l'Union européenne réagisse et s'engage, elle aussi a privilégié des achats européens le commissaire européen français Thierry Breton, appelle à la création d'un fonds européen de souveraineté pour soutenir des projets industriels. Ce projet sera-t-il évoqué au Conseil européen. La question des relations transatlantiques figure en effet à son ordre du jour mais nous savons aussi que certains outre-Rhin jugent propice le moment pour relancer les négociations d'un accord de libre-échange entre l'Union et les États-Unis. Pouvez-vous nous rassurer à cet égard Madame la Ministre je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Dans la suite du débat. La parole est aux orateurs des groupes. Et nous allons entendre Madame Véronique Guillotin groupe Rassemblement démocratique et social européen pour six minutes, chers collègues. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis le début de l'année la question de l'Ukraine occupe naturellement une grande partie de l'ordre du jour des conseils européens qui se succèdent. Nous aurions aimé qu'il en soit autrement. Hélas, la poursuite de l'agression russe intensifié par des frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes pousse repousse chaque jour l'espoir d'un retour rapide à la paix. Cette situation dramatique aux portes de l'Europe nous conduit à rester encore au chevet de l'Ukraine. La lassitude ne doit pas l'emporter sur notre engagement en faveur de la liberté de nos amis ukrainiens d'autant moins qu'il s'agit aussi de protéger la nôtre à plusieurs reprises jusque sur les bancs de l'ONU en septembre dernier, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Vladimir Poutine a clairement déclaré la guerre aux valeurs démocratiques défendus par l'Occident. Alors oui quel que soit le coût de cet engagement mon groupe soutient toutes les initiatives menées d'un côté pour sanctionner la Russie et de l'autre pour apporter des solutions militaire et humanitaire à Kiev. Nous approuvons en effet les différents leviers utilisés jusque là pour aider l'Ukraine, que ce soit l'assistance macrofinancière exceptionnelle de 9 milliards d'euros acté par le Conseil du 20 septembre dernier l'aide d'urgence humanitaire ou encore la mobilisation de la Facilité européenne pour la paix. En tant que présidente du groupe d'amitié France-Moldavie, je me réjouis également de l'attention particulière portée à ce pays et certains de ses voisins. Le chef de l'État l'a rappelé il y a 2 semaines aux côtés de la Première ministre moldave lutter pour la Moldavie c'est participer à l'effort de guerre que nous conduisons aux côtés de l'Ukraine. Nous savons bien que la déroute des troupes russes en Ukraine épargne pour le moment les projets à peine voilée de Moscou en Transnistrie. La communauté internationale doit donc demeurer vigilante. S'agissant du soutien qui FINA ou entre les dons, les prêts et les projets financiers avez-vous madame la ministre, une évaluation du montant cumulé des aides à la Moldavie.-- En ce qui concerne les sanctions contre Moscou. Il faut espérer que la dernière mesure, celle de l'embargo sur le pétrole brut russe. Entré en vigueur hier rempli son objectif de tarissement du financement de la guerre. En revanche, il est certain que le dispositif de plafonnement du prix du baril pour ceux qui continueront à importer du pétrole russe constitue une brèche. On peut le regretter, mais il est important de ne pas déstabiliser le marché mondial, plus qu'il ne l'est déjà. Il s'agit aussi de ne pas alourdir outre mesure le choc énergétique qui fragilise déjà beaucoup les économies européennes à cet égard qu'elle accueille. La France va-t-elle réservé au projet de compromis relatifs au mécanisme de correction du marché des prix du gaz récemment avancée par la présidence tchèque. Il existe une ligne de fracture au sein de l'Union européenne, qu'il faudra bien finir par aplanir pour avancer. Les conclusions du Conseil européen des 20 et 21 octobre demande un nouvel indice de référencement qui reflètent plus exactement les conditions du marché du gaz. Il est urgent de les mettre en oeuvre en 2023. Le temps presse. En effet face à une inflation qui qui relativise les efforts des États en matière d'action publique qui soit pour les ménages, les collectivités locales, les entreprises de bouclier tarifaire de l'électricité et du gaz est un outil opportun dans cette période où il est demandé de faire preuve de résilience. Il est fondamental de protéger les plus vulnérables de l'inflation, mais jusqu'à quand nos finances publiques vont elles permettent de tenir ce cap en outre un véritable chapitre social cohérent reste à ouvrir en Europe. Si la guerre en Ukraine a précipité le défi énergétique, il apparaît clairement que la sobriété risque de durer. Compte tenu de l'accélération avérés du réchauffement climatique dans ces conditions, nous attendons une réponse globale et stratégique de long terme, porter à 40% l'objectif de l'Union européenne en part d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique d'ici 2030, soit 8 points de plus que la cible en vigueur est une nécessité. J'espère que les trilogues aboutiront à ce niveau. qui représente un compromis acceptable pour notre pays qui, disons-le, accuse un retard en matière d'énergies renouvelables enfin sa thèse à cette crise et la récession qu'elle entraîne l'Union européenne, sans renier les règles de l'OMC doit par ailleurs s'affirmer face à certaines initiatives de ses partenaires peu respectueuse des règles du jeu. Je pense aux femmes hier à du président Joe Biden. Ce plan de 420 milliards de dollars qui contient une part de subventions et de réduction d'impôt est-il de nature à créer une exode massive de nos industries outre-Atlantique comme on l'entend. Quel est le résultat du conseil ministériel du commerce et des technologies entre les États-Unis et l'Union européenne sur ce sujet. Mon groupe n'est pas partisan d'alimenter un conflit commercial ou d'appeler au protectionnisme en représailles. Cependant, nous attendons de savoir quelle réponse systémique entend mettre en oeuvre. Bruxelles pour protéger les entreprises européennes Il me semble qu'il serait souhaitable d'encourager la délivrance des agréments pour les projets d'intérêt européen d'une part et de revoir le cadre des appels d'offres publics d'autre part. Mes chers collègues. Sans transition, je souhaiterais terminer sur l'Europe de la santé un peu relégué à l'arrière-plan alors que l'épidémie de Covid, n'a pas disparu. Où en sommes-nous. Madame la Ministre du paquet pour l'union de la santé. La commission devrait notamment remettre en début d'année sa proposition de législation générale européenne concernant les médicaments mon groupe sera particulièrement attentif aux problématiques d'accès aux médicaments, ainsi qu'aux levier pour une industrie pharmaceutique innovante et leader en Europe. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pascal Alizart pour le groupe Les Républicains et pour six minutes. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, l'année 2022 remarquer le retour de la guerre sur le continent européen il y a Total, qui vise autant l'armée ukrainienne que les populations. Pour l'instant les desseins du président russe annexer l'Ukraine y installer son pouvoir diviser et affaiblir les Européens ont été mis en échec. Cet événement géopolitique majeur a forcé l'Europe agir, réagir avec fermeté et unité. La mise en oeuvre du Fonds européen de défense, l'adoption de la boussole stratégique, la volonté d'accroître l'effort de défense et de mutualiser les achats militaires vont indéniablement dans le bon sens. Malgré les mesures prises et l'unité affichée des Européens. Nous sommes en réalité encore bien fragile face aux soubresauts du monde à l'affirmation de puissance désinhibée à la dégradation du système multilatéral. Les sanctions européennes n'ont pas permis pour l'instant d'affaiblir le pouvoir et l'économie russe autant qu'espéré. Depuis plusieurs mois les vendredi trop d'hydrocarbures russes à la Chine sont en hausse et permettent en partie de pallier la défection des Occidentaux. Une Russie très affaiblie voire exangue est dépendante de la Chine ne me semble pas à terme une bonne perspective pour la sécurité de l'Europe et pourtant ces sanctions sont nécessaires. Le bannissement des production pétrolière et gazière russe conduit à une crise énergétique déstabilisante. Elle a mis en lumière la dépendance et la légèreté de certains États membres en matière d'approvisionnement. Par ricochet, la filière nucléaire revient en grâce. Mais après avoir été durablement affaibli et dénigrer nous risquons ainsi des coupures de courant cet hiver. Factuellement, la recherche de solutions alternatives ne va-t-elle pas conduire à de nouvelles dépendances Gaz de schiste américain production du Golfe ou de la Caspienne avec les conséquences géopolitiques qui en découlent. Le projet re-Power il European Yonyon sera-t-il adapté et constitue-t-il vraiment une opportunité pour la France. Ces évolutions en matière de sécurité, d'énergie de souveraineté seront-elles pérenne et avec le temps Madame la Ministre ne risque-t-on pas de revenir au Business as Young as Usual au détriment d'une vision stratégique global. Enfin, cet intérêt nouveau des Européens pour la défense profite surtout à la résurrection de l'OTAN et se manifeste largement par l'achat d'équipements militaires structurant américain. L'BIT D européenne doit être privilégié les coopérations rechercher chaque fois que cela est possible sans s'interdire des développements strictement nationaux lorsque des coopérations s'avère préjudiciable à nos intérêts. Parmi les autres points d'inquiétude. Je rappelle les mesures protectionnistes américaines, dont les plus récentes. L'inflation réduction Act prévoit près de 400 milliards de dollars d'aide à la relou que les la relocalisation pardon sur le sol américain d'industrie d'avenir. Il y a là une menace directe pour l'Europe et je partage tant les propos du président de la commission des Affaires européennes que ceux de l'oratrice précédente. Le commissaire, Thierry Breton, appelle à la création d'un fonds européen de souveraineté. Qu'en est-il réellement Madame la Ministre concernant la Chine une prise de conscience commencent à émerger au niveau européen. À propos du déséquilibre des échanges du non respect de la propriété intellectuelle des différences de normes sociales et environnementales ou de ses visées géopolitiques pour autant des projets de cession d'infrastructures européenne à des entreprises chinoises demeure. N'aurions-nous pas retenu la leçon du Pirée. Nos voisins britanniques viennent d'évincer un actionnaire chinois de leur principal fabricant de semi-conducteurs et d'interdire l'installation de caméras produites en Chine pour la visio surveillance des sites sensibles. Par ailleurs, où en est le projet Global Gateway qui se voulait une alternative tueuse à la BRI chinoise n'est-il pas trop contraignant. Face à une offre chinoise qui s'adapte en fait aux réalités locales, sur les côtes de la Manche, la pression migratoire s'est fortement actually accentué pardon en 2022. Les Britanniques vont augmenter leurs versements à la France pour enrayer les traversées mais du fait lors économie continue d'absorber ces flux de migrants illégaux. L'effet d'attraction demeure on fustige certes l'attitude du gouvernement italien dans l'affaire de l'Océan Viking. Mais c'est précisément la question migratoire non résolu les 100 parfois l'Italie bien seul. Qui est l'une des causes majeures de l'arrivée au pouvoir de cette majorité populiste et cela pourrait bien arriver ailleurs si des mesures plus fermes ne sont pas prises. Enfin Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur la situation en Birmanie. Ça peut sembler loin de l'Europe mais l'exécution de 11 jeunes étudiants par la junte est prévue pour demain. C'est totalement inacceptable. Madame la ministre, où sont les protestations françaises et européennes. Le prochain conseil européen devrait, me semble-t-il aussi prendre position sur ce sujet. Voilà. Madame la Ministre, mes chers collègues, madame la présidente, les quelques observations que je souhaitais partager avec vous avant ce conseil européen. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Pierre mais de vielles pour le groupe les indépendants et pour six minutes.

Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. À la lumière du contexte international de la guerre en Ukraine mais également de l'urgence climatique. Le prochain conseil européen devant nous permettre. De proposer des solutions pour faire baisser le prix de l'énergie. D'évoquer la défense et la sécurité européenne. Mais également, de renforcer nos relations avec nos voisins des Balkans. Tout d'abord, c'est bien la question énergétique qui aujourd'hui nous préoccupe en 1er lieu. En effet, l'Europe qui dépendaient jusqu'alors des hydrocarbures russes, se trouve aujourd'hui dans une situation difficile. Ce qui annonce un hiver particulièrement complexe. Il nous faut trouver une réponse collectivement.-- J'insiste sur le mot collectivement car si nous prenons l'exemple. Du prix de l'électricité et de sa connexion auprès du Il n'est pas aisé de trouver une solution qui puisse satisfaire tout le pays. Étant donné la diversité des degrés de dépendance, on est aux énergies fossiles. Les actions solitaires qui pourrait à terme déstabiliser l'Union sont à écarter.-- C'est bien sur le volet énergétique. Que nos désaccords sont le plus profond. À l'image du du rendez-vous manqué entre les ministres européens de l'énergie. Il y a des jours sur le plafonnement du prix du gaz. Madame la Ministre quelles sont vos lignes rouges et vos espoirs pour faire avancer ce dossier la semaine prochaine.-- L'urgence est également d'actualité en termes de défense.-- Vous expliquez récemment Madame la Ministre que nous entrions dans une nouvelle phase des relations franco-allemandes. Force est de constater que les coopérations reste longue et parfois difficile. J'en profite pour vous interroger, tout particulièrement sur le projet du système de combat aérien. Le Scaf lancé déjà depuis 2017. Et qui peine avancer. Comme chacun le sait, les négociations ont pris un sérieux retard. Et cette situation dessert de plus en plus. La préparation nos nos armées à la guerre aérienne du futur.-- Je me réjouis cependant de voir que nos deux pays avant sur le sujet et que Dassault Airbus poursuivent leur collaboration.-- À ce titre, pouvez-vous nous en dire davantage sur des avancées concrètes. Suite à l'accord européen sur le démarrage de la phase 1 B d'étude du démonstrateur annoncé par le gouvernement allemand le 18 novembre 2022.-- Notre stratégie en termes de défense implique une industrie d'armement militaire forte. Et l'achat de produits européens. Nous ne pouvons que déplorer les commandes de F-35 américain passer par les Allemands.-- Lors de la rencontre une autre combien bien administre avec le chancelier allemand qu'est-il ressorti des discussions sur le volet défense. Il était aussi question d'un Mbaye European Act quelles évolution attendons-nous. Au-delà de ces questionnements notre position européenne sur le conflit en Ukraine et clair. Je tiens notamment a salué le vote de la proposition de résolution sur la reconnaissance de la Fédération de Russie en tant qu'État soutenant le terrorisme. Cette résolution condamne bien sûr la Russie de Poutine. Et réaffirmons notre soutien aux Ukrainiens. Je le rappelle ce soutien prendre diverses formes. Et nous, au nord. Nous devons poursuivre sans relâche nos efforts. La résolution ont été établis pardon plusieurs demandes en direction de la Commission européenne et des États. L'une d'entre elles concernent la création de mécanisme mondial. De sanctions contre la corruption. Quelle est la position de la France sur ce sujet. Enfin je souhaite évoquer nos relations avec les pays des Balkans. Le sommet qui s'est tenu aujourd'hui à Tirana. Et l'occasion pour les européennes de réaffirmer leur engagement dans la région. De reconfirmer les avancées progressives d'adhésion des Balkans occidentaux. Et d'appeler à l'accélération des négociations. En octobre dernier. La commission a notamment recommandé d'octroyer le statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine. Cette décision reviendra au Conseil européen des 15 et 16 décembre. Ce lien. On avait les Balkans occidentaux et d'autant plus nécessaire en raison de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Cette guerre aux portes de l'Europe nous oblige à renforcer rapidement de nos décisions, à 27. Nous ne pouvons pas reporter indéfiniment nos choix commun. Différentes dossiers restent dans l'impasse et particulièrement le découplage des prix de l'électricité et du gaz.-- Le Conseil européen. Doit réussir le chemin à trouver son chemin pour répondre à notre défi énergétique. Il sera décisif. Soyez assurée Madame le Ministre notre soutien, enfin je pense qu'il faudra aller au-delà d'une réponse structurelle, basée sur le marché de l'énergie. Cette crise dont nous emmenaient plus loin nous devons revoir nos modes de vie et de consommation. Ne pas revenir. Ne pas revenir à la bougie ou la lampe à huile, comme le réclament certains prédicateurs ni tomber dans la radicalité mais nous devons nous adapter grâce à l'innovation et à l'Intelligence collective. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jacques Fernique. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour six minutes.

A une détermination commune sans précédent pour soutenir l'Ukraine. Il s'agit en effet d'une attaque contre nous tous contre nos valeurs communes contre les chances aussi du multilatéralisme pour changer la donne planétaire, c'est aussi d'une certaine façon là le défi du climat qui se joue un peu en Ukraine. Face à une situation inédite des des décisions impossible il y a encore quelques mois ont été prises en quelques semaines, renforçant l'évidence ce n'est qu'ensemble que les États membres de l'Union auront le poids suffisant face à la crise énergétique, les États n'ont pas tous la même capacité à gérer équitablement les prix et la demande ou à fournir le soutien est essentiel à ceux qui en ont besoin. La solidarité européenne est donc essentiel ce Conseil européen doit permettre réforme vers la réponse commune. Aux enjeux des coûts et des approvisionnements énergétiques, une réponse commune qui soit abouti crédibles, pertinentes pour reprendre vos adjectifs et ceux du président Rapin hein il y a un instant. Cette réponse aboutit elle sera cohérente avec nos objectifs climatiques si elle contribue à la réduction de notre dépendance à l'égard des importations d'énergies fossiles. Et des combustibles fossiles en général en particulier avec des régimes autoritaires. Je crois que la stratégie à court terme favorisant de nouveaux investissements dans des pays tiers comme l'Azerbaïdjan ne va pas dans ce sens. Face à la réponse états-unienne à la crise avec leur bas prix de l'énergie avec leur plan massif de centaines de milliards de dollars de l'inflation réduction Act orienter résolument vers la transition et la décarbonation industriel notre Green Deal européen risque fort de faire pâle figure la compétitivité de nos économies se joue dans ce défi. La fragmentation de nos économies européennes est un péril imminent. Oui un nouvel élan européen est nécessaire, il nécessite de trouver les voies. Pas facile d'un accord pour un plan massif qui soit d'une certaine façon une amplification industriel du Green Deal. Avec des investissements à la hauteur et donc. Pour constituer ce fonds de souveraineté un emprunt commun nouveau ce nouvel élan européen nécessite de hâter la mise en place concrète de l'ajustement carbone aux frontières. Ce. Protectionnisme Vert européen ce juste échange, si on préfère qui équilibrera notamment la relation avec la politique américaine, c'est la volonté de protéger nos économies en transition de concurrents qui méprisent l'environnement, le climat, les droits sociaux, les droits humains. Or, le Conseil a adopté jeudi dernier sa position sur la directive devoir de vigilance et on ne peut pas dire que notre gouvernement français et jouer un rôle positif. Le secteur financier et de facto dégager de toute responsabilité. Oui, le gouvernement français champions du devoir de vigilance dans ses discours a d'une certaine façon affaiblit l'ambition du projet de directive européenne la semaine passée, il a entraîné avec lui, l'Espagne, l'Italie. Pour rappel, les banques françaises ont investi plus de 743 millions d'euros dans la déforestation du Brésil, on ne peut pas ainsi les exempté de toute responsabilité. Avec la loi sur le devoir de vigilance dans le détail, votre gouvernement a poussé au conseil pour que les mesures d'évaluation et de prévention des risques. Demander aux entreprises ne soient que volontaires pour les banques. Or, sans obligation, pas d'action, les banques pourraient donc continuer comme BNP Paribas qui est le 1er financeur des fossiles en Europe. Pourtant la France était le 1er pays en 2017 à avoir inscrit dans son droit le devoir de vigilance qu'est devenu notre rôle de leader européen pour défendre des ambitions élevées pour les droits humains et l'environnement. Mais les lobbies ont du talent. Les intérêts sont ailleurs. Le texte adopté au Conseil et décevant il exclut la possibilité pour des victimes. D'agir en justice pour être indemnisés. Lorsque l'entreprise a manqué à ses obligations environnementales, le climat a également été exclu du texte final tandis que les dommages environnementaux en général devront être identifiés mais sans engager aucune responsabilité. Aurons-nous une loi d'apparence, pour reprendre les mots de Dominique Potier. Le père de notre loi pionnière française. n'a peut-être pas dit son dernier mot. Espérons qu'il pourra peser comme il l'a fait pour l'accord historique de la nuit dernière pour protéger les forêts du monde et garantir aux Européens des paniers de courses sans déforestation en imposant aux entreprises, ce qui est un devoir de vigilance sur la déforestation liées à leurs activités, c'est sur 16% de la déforestation mondiale dont l'Europe et responsable que nous agirons des ambitions élevées ont été maintenus en incluant le caoutchouc le charbon les dérivées de l'huile de palme. Certes, le secteur financier à un peu réussi son lobbying pour être exclu dans un 1er temps du règlement. On y reviendra dans 2 ans. Une ambition politique du même ordre devrait animer le conseil pour que le fonds social pour le climat évite la casse sociale des transitions nécessaires, l'abandon pur et simple de l'extension du marché carbone. Ah la route et au bâtiment serait désastreux de ce temps de ce point de vue oui, il faut éviter de taxer les ménages populaires mais les usages commerciaux peuvent et doivent l'être le dernier trilogues n'a permis aucune avancée. Nous comptons sur une action résolue pour y parvenir. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles aboutir vite sur une politique d'approvisionnement et de coûts énergétiques partagé porter le Green Deal au niveau qui s'impose, ne pas renoncer ni sur la vigilance des entreprises ni sur le fond social pour le climat. Autant d'ambition pour le nouvel élan européen. Nécessaire. Merci cher collègue. La parole est à monsieur André Gattolin groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour 9 minutes, chers collègues. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues lors du précédent débat préalable en octobre dernier. J'avais déjà eu l'occasion de souligner que jamais jusqu'à l'heure, l'ordre du jour de conseil n'avait été autant porter sur des thématiques internationales internationales et géostratégique alors dans mon enthousiasme d'Européen convaincu, je voulais lire là les prémices d'un possible réveil géopolitique de l'Europe. Il ne saurait en effet y avoir d'union solide et pérenne. Sans un tel réveille. Et je le répète qui est à l'AC je là souvent jamais au cours de l'histoire un regroupement volontaire d'Aida d'État démocratique ne s'est constituée autrement qu'à la suite d'une confrontation politique et militaire majeur qu'il s'agisse d'une guerre d'indépendance d'une guerre civile d'une guerre de libération ou encore d'un conflit d'ampleur avec une puissance extérieure agressive alors. L'Union européenne serait-elle en la matière une divine exception. On l'oublie parfois, mais ce sont pourtant bien des préoccupations géopolitiques qui ont été au coeur des premiers pas de la construction européenne, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la création d'abord du Conseil de l'Europe en 1949 puis celle de la CECA en 1951, je le rappelle, le 1er marché européen de matières premières stratégiques à travers le charbon et l'acier et même limités dans leur périmètre ces 2 exemples illustrent bien mais patatras en 1954 avec l'échec de la Communauté européenne de défense et le repli contraint des pères fondateurs de l'Europe, sur une distance dimension. Plus strictement économique de la construction européenne. L'infâme agression russe contre l'Ukraine et ses multiples conséquences remettent aujourd'hui. Cet enjeu géopolitique au centre du village Europe. l'ordre du jour prévu. Notionnel de ce Conseil des 15 et 16 décembre prochain avec cette fois-ci pas moins de 6. Ayant tous une portée géopolitique et géostratégique indéniable. Poser les bonnes questions s'est dit ont déjà commencé d'y répondre et il faut le reconnaître. Depuis janvier dernier de surtout février dernier jamais l'union n'aura 80 avancer tant en matière d'Europe de la défense d'union des marchés de l'énergie que de lutte contre les ingérences étrangères. étrangères. Sans vouloir être rabat-joie, je rappellerai cependant que le verre à moitié rempli nos cure pas nécessairement du fait qu'il sera plein un jour dans ce type de débat et les fréquences sans le lire d'ailleurs de citer Jean Monnet quand il écrivit que l'Europe se ferait dans les crises et quelle serait la somme des solutions qu'on apporterait à ces crises, c'est vrai, mais on oublie en général de rappeler que toutes les crises traversées par l'Europe n'ont pas fait systématiquement l'objet d'une réponse adéquate et que par ailleurs l'essentiel des crises affronter par l'Union depuis les années 60 étaient des crises de nature économique et financière et que les réponses apportées venait de fait renforcer encore la nature essentiellement économique et commercial de l'Union jusqu'à présent les moments géopolitique. Cruciaux donc que rarement fait l'objet de réponse européenne à la hauteur des enjeux. À la suite de la chute du mur de Berlin, puis de l'effondrement de l'URSS, l'Union a certes réagi en acceptant la réunification de l'Allemagne et en procédant un très vaste élargissement incluant les pays libérés du joug soviétique, mais nous avons renoncé à l'époque à nous doter d'une gouvernance politique renforcée et surtout d'un système de défense propres à l'Europe qui aurait véritablement consolider notre réponse. Je m'agace aussi quand j'entends dire que l'actuelle guerre en Ukraine marquerait le retour de la guerre sur le territoire européen. Après 70 années de paix, c'est faire en effet bien peu de cas de la succession de conflits sanglants qui se déroulèrent dans les Balkans occidentaux entre 1991 et 2001 et qui causa la mort de plus de 140.000 personnes. Il faut dire que la réponse de l'Union à l'époque n'a pas été à la hauteur et que ce sont les États-Unis et l'OTAN, qui ont été à l'époque les maîtres d'Oeuvres désengagement militaire visant à mettre fin à ce conflit. Alors oui, dans la guerre en cours. Les pays européens ont franchi un pas très significatif mais un pas qui reste d'importance mais un effet inférieur à celui effectué par les États-Unis précisément dans ce conflit et je m'interroge parfois de savoir si notre engagement eut été le même si Washington n'avait pas fait le choix qui est le sien depuis plus de 9 mois et pour reprendre Jean Monnet je dirais que c'est la somme des réponses que nous apporterons aux crises géopolitiques qui nous frappe qui permettra de dire sur le l'Union européenne est véritablement en train de franchir une étape décisive ou si au contraire une fois le conflit passé, nous ne nous laisserons glisser à nouveau vers le Business as Usual pour ne céder pour ne pas céder à une indifférence qui confine Real à l'acheter. Nous devons garder je crois sans cesse à l'esprit le courage et la détermination des Ukrainiens qui nous rappellent tous les jours que la liberté n'est pas une option que c'est un combat à ceux qui aujourd'hui jouent Pékin en pensant que Xi Jinping pourrait convaincre Vladimir Poutine d'arrêter sa guerre sanglante contre les Ukrainiens. Je dis qu'ils connaissent très mal les actuels dirigeants de la Chine et de la Russie. Et si à force d'exactions et de crimes de guerre commis par la Russie. Les Européens se positionne tu enfin clairement par rapport à Vladimir Poutine. Il est loin d'en être de même vis-à-vis de Xi Jinping et de son pouvoir ultra-autoritaire et de plus en plus ouvertement expansionnistes lors de la dernière réunion du Conseil européen. Nos chefs d'État et de gouvernement se sont bien poser la question de l'évolution de leur positionnement face à la nouvelle équation chinoise mais là encore, nous sentons une vraie fille frilosité à mettre clairement des mots sur les choses puisque ce débat a eu lieu dans un cas dans le cadre d'un point, vraiment très sobrement intitulé dans l'ordre du jour, relations internationales. Et. Comme par hasard. Bis répétita pour le Conseil à venir point 2. Référant explicitement à la Chine. Pourtant, on ne voit guère comment ce sommet qui se tiendra je le rappelle au lendemain d'un sommet Union européenne-Asie Hazem et Asean à Bruxelles et surtout quelques jours après les soulèvements inédit, qui se sont produits contre la folle politique de zéro Covid des autorités chinois. Je ne vois gare guerre comment le Conseil n'en parlerai pas. Alors je le dis c'est en osant enfin nommer les choses par leur nom que notre union pourra véritablement affirmer son virage géopolitique. Un virage aujourd'hui indispensable à son existence pleine et entière, voire même à sa survie dans un monde où la brutalisation des relations internationales, n'est plus une menace mais bel et bien une réalité. Je vous remercie. Merci cher collègue hein. La parole est à monsieur Didier Marie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Pour sept minutes.--

Madame la présidente Madame la Ministre, chers collègues. Le Conseil européen des du 15 décembre vient clore une année qui aura profondément bouleversé l'Europe. Confronté à la guerre à ses portes, l'Union à surréagir se montrer unis comme Janet, mais a aussi vu ses faiblesses mises à nu. Solidaire, d'abord avec l'Ukraine sur le plan financier avec le déblocage de 18 milliards d'euros. Madame la Ministre la rappeler. Solidaire sur le plan militaire, avec les 3 milliards de l'instrument de facilités pour la paix qui ont permis de livraison massive d'armes qui, ajouté au courage des Ukrainiens, a permis dans un 1er temps de résister à l'offensive russe, puis de contre-attaquer avec succès. Solidarité humanitaire avec la mise en oeuvre pour la première fois de la protection temporaire, qui vient d'être allongé jusqu'en mars 2024 et a permis l'accueil de plusieurs millions de réfugiés dont 100.000 en France. Solidarité enfin pour sanctionner la Russie même s'il aura fallu discuter et que l'on pourrait vraisemblablement aller plus loin. Tout cela est à saluer, et l'Europe doit rester unie et déterminée dans son soutien à l'Ukraine et la condamnation sans concession de l'agresseur qui est la Russie. Permettez-moi, à cet instant Madame la Ministre, de vous dire mon étonnement d'avoir entendu le président de la République aborder la nécessité de donner à monsieur Poutine, je cite, des garanties de sécurité alors que lui ne donne aucun signe de désescalade, bien au contraire, en transformant l'hiver en arme de guerre contre les civils en détruisant impitoyablement les infrastructures énergétiques du pays.-- Ce n'est à nos yeux ni à nous ni le moment de tendre la main.-- Si l'Union a su réagir la guerre marque cependant un avant et un après pour l'Europe. Nos certitudes s'évanouissent. L'Union européenne n'est plus protégé. Elle ne peut se défendre au sol et des l'ex-sa sécurité au parapluie militaire américain. Sa prospérité fondée sur la pérennité de la paix est ébranlée comme son économie qui se posait jusqu'à présent sur une énergie bon marché. L'inflation s'installe la récession menace la crise énergétique frappe les ménages et fragilisent notre tissu industriel. Notre démocratie elle même vacille sous la désinformation les ingérences étrangères et la montée des populismes comme nous l'avons amèrement constaté en Suède et en Italie. L'Europe doit faire front conforter son unité et ne pas céder à la fragmentation. Nous devons assumer nos responsabilités reconstruire nos souverainetés réduire nos dépendances. Cela commence dans l'urgence par des réponses à la crise énergétique. Les divergences entre États nous font perdre un temps précieux. Si un accord a pu être trouvé sur le pétrole russe, qu'il faut aller plus loin et conclure sur l'achat de gaz en commun, créer un fonds européen de soutien aux ménages et aux entreprises découpler le prix de l'électricité, celui du gaz. C'est une priorité absolue et nous espérons que le récent rapprochement des points de vue entre la France et l'Allemagne pour une réforme structurelle du marché de l'électricité permettra d'aboutir très rapidement et évitera la menace de délocalisations de nos industries. Ensuite viendra le temps de bâtir notre indépendance énergétique. En investissant massivement dans les énergies renouvelables en évitant qu'une nouvelle dépendance au gaz de schiste américain cher ou à l'Azerbaïdjan ne succède à celle que nous avions avec la Russie. Se posera aussi la sécurité de nos approvisionnements en matières premières l'uranium par exemple aujourd'hui importés de pays peu sûrs et dont les déchets sont recyclés en Russie, seul pays habilité est en mesure de le faire. 2ème point d'urgence l'inflation à 11 et demi pour 100 en moyenne européenne, en octobre dernier elle fait crainte de réels risques de récession. À ce sujet le relèvement des taux d'intérêt par la BCE fait émerger de nombreuses inquiétudes notamment pour l'accès au crédit. Cette situation pose aussi la question de notre politique budgétaire et celle de la reconduite ou non du pacte de stabilité. Pouvez-vous Madame la Ministre de nous éclairer sur la position que la France défend. Pour éviter la récession. Bâtir notre autonomie stratégique relever les grands défis climatiques et industriels. L'Europe doit investir. Pouvez-vous nous préciser la position du gouvernement sur la faisabilité de lever un grand emprunt communautaire pour financer ses investissements. Alors que le ministre allemand des Finances ne lui apporte manifestement pas son soutien. Cette guerre nous affaiblit après un épisode sanitaire qui avait déjà souligné nos dépendances et dans un contexte de tensions croissantes entre les USA et la Chine. Nous devons à la fois renforcer notre politique industrielle commune. Continuer d'agir pour réduire nos dépendances rester solidaires et porter nos valeurs dans le contexte international. À cet égard les récents déplacement d'Olaf Scholz puis de Charles Michel à Pékin et celui du président Macron aux USA semble s'inscrire dans une volonté de porter la voix économique et commercial de l'Union européenne face à de puissants certes différentes mais qui n'ont ni l'une ni l'autre d'état d'âme. Mais les objectifs de l'Allemagne sont-il bien compatible avec ceux du reste de l'Union européenne. L'état des relations franco-allemandes a suscité de nombreuses réactions. Ces dernières semaines. Pouvez-vous Madame la Ministre, nous faire un point sur les convergences et les divergences entre nos 2 pays. Prévoyez-vous un nouveau conseil des ministres commun après l'annulation de la première initiative.-- Le président de la République lors de sa visite d'État aux États-Unis a pointé le danger que représenterait l'inflation dans la réduction Act et ses 370 milliards de subventions et allégements fiscaux aux entreprises américaines engagées dans la transition vers une économie décarbonée. Très bien. Mais ne soyons pas naïfs, les Américains ne nous épargneront pas. Nous devons bien évidemment de négocier, mais parallèlement nous protéger. Alors Madame la Ministre à quand un Bayou European Act comme le demande le Parlement européen depuis de nombreuses années. Enfin cette guerre aux portes de l'Europe nous interroge sur le positionnement géostratégique de l'Union européenne et de ses relations de voisinage. La question de l'élargissement est ainsi revenu sur le devant de la scène. Il est temps de mettre en oeuvre une méthodologie clarifier et harmoniser pour accélérer les négociations répondre à l'envie d'Europe des peuples des Balkans occidentaux de l'Ukraine et de la Moldavie et de freiner l'influence croissante. De puissances étrangères qui déstabilisent ces pays. Le sommet UE-Balkans qui a lieu aujourd'hui et le soutien d'un milliard d'euros pour faire face à la crise énergétique sont les bienvenus mais il faut donner des gages supplémentaires à ces pays tout en conservant à haut niveau d'exigence vis-à-vis des règles européennes. Pour conclure après 6 mois de présidence française et 6 mois de présidence tchèque cette année 2022 aura permis certaines avancées, notamment sur la solidarité des 27 à l'égard de l'Ukraine. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Il est temps de passer de la parole aux actes pour construire une Europe plus puissante plus résilientes et plus ambitieuse. La France doit jouer un rôle moteur dans cette transformation. Madame la Ministre, nous souhaitons que le président de la République et vous-même fassiez preuve de diplomatie de conviction et de fermeté lors de ce Conseil européen pour enfants engager des avancées sur les dons aux sujets évoqués aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur le président, Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 7 minutes.

Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues. Nous débattons ce soir à la veille d'un Conseil européen qui se tient dans un contexte d'aggravation certaine en 2023 de la crise énergétique économique au sein de l'Union.-- Toute une partie de la zone euro et menacé d'entrer en récession en 2023. Et selon les estimations de la Commission européenne, les gouvernements de la zone euro. Jusqu'à présent consacré déjà collectivement environ 1,25 du PIB intra-zone au soutien à l'énergie, ce qui représente déjà environ 200 milliards d'euros. En France, nous sommes aujourd'hui face à des prix qui ont dépassé 1000 euros le mégawattheure cet été et qui sont aujourd'hui aux alentours de 500 ou 600 euros le mégawattheure, soit une multiplication par 10 à 20 par rapport au prix d'avant crise sanitaire. Si cette hausse a été exacerbée par la crise ukrainienne. Il est admis que ces prémices sont antérieurs. Dès juillet 2021, les tarifs réglementés de l'électricité en France ont connu une envolée vertigineuse du fait d'un emballement des prix sur le marché de gros. Les prix de gros du gaz ont augmenté de 150% entre avril 2021 et fin octobre 2021. Pour un client moyen, la facture de gaz est passé de 977 euros à 1492 euros. Par conséquent, le prix de l'électricité sur les marchés de gros corrélé au prix du gaz a été complètement détourné des coûts de production avec un triplement des prix en un an l'électricité nucléaire française a connu alors une décorrélation de ses coûts de production et de sa valeur sur les marchés. C'est vrai qu'en 2022 l'augmentation des coûts de production a été importante du faire de, du fait de l'indisponibilité d'une partie de notre parc nucléaire. La sécheresse a aussi eu un impact sur le volume de production hydroélectrique toutefois nos coûts de production sont restés très inférieur au prix de marché. Je prends soin de faire ce rappel car la crise ukrainienne ou le manque de capacité de production, en particulier en France n'explique pas la spirale haussière le faire serait passé à côté des véritables enjeux, la crise énergétique n'est pas conjoncturelle elle est structurelle. Elle tient à l'organisation même du marché de l'énergie celui l'électricité en particulier il faut bien constater que c'est la part mineure de l'énergie, échanger sur le marché de gros, qui nous entraîne dans cette spirale inflationniste qui met aujourd'hui en danger. Les particuliers, les collectivités et les entreprises. Cette fragilité du marché unique européen de l'énergie est aujourd'hui largement documenté la France répète à qui veut l'entendre depuis des mois qu'il faut sortir du mécanisme de la dernière centrale appelée mais devant les refus catégorique notamment de l'Allemagne, on se borne pour le moment à constater les dégâts. Le plafonnement de la ronde des infra-marginaux à 180 euros le mégawattheure, soit au minimum trois à quatre fois leurs coûts de production continuerait de tirer les prix à la hausse en France, en maintenant d'énormes profits pour ses producteurs aux dépens des consommateurs et des contribuables. Tout porte à croire que les mécanismes proposé d'ailleurs très complexe n'ont pas été suffisamment étudiés qu'ils sont, au mieux, inefficaces au pire contreproductif. Et qu'ils laisseront la place à de nombreux effets de domaines comme ceux liés à la reine ou dernièrement à la sortie de l'obligation d'achat et la promotion des power purchase agrément de ces contrats privés bilatéraux avec un droit de tirage de soutirage pour les acteurs privés. Imaginez pour favoriser les investissements de long terme devant la faillite des effets spéculatifs du marché revient de fait à accepter de confier les moyens de production à des grands groupes privés français ou étrangers. Et dans ces conditions, la décentralisation des moyens de production mais aussi l'éclatement du réseau distribution porte en germe les risques d'une remise en cause de la péréquation tarifaire de l'électrique du prix de l'électricité et de l'égalité territoriale les solutions consistant à se défaire de ce prix de marché pourtant largement responsable de la crise sont pour le moment éliminé d'office car contraire au dogme de la concurrence. Mais madame la mini-c'est bien pourtant cette réforme en profondeur du marché européen d'électricité que la France doit porter et sur laquelle nous venons de déposer une proposition de résolution elle doit articuler des mesures immédiates, comme l'extension des tarifs régulés, comme nous le proposons demain dans notre espace réservé pour les collectivités locales, la négociation de dérogations permettant à la France de rapprocher les prix nos coûts de production, compte tenu de la spécificité nucléaire de notre mix et le plus vite possible, possible avancer vers une exclusion l'électricité des mécanismes concurrentiels, à commencer par une décorrélation des prix de l'électricité et du gaz. C'est urgent, d'autant que les mécanismes de soutien compenser les folies du marché coûte très cher. Le seul bouclier tarifaire en France, a estimé après déjà de 45 milliards d'euros.-- Je voudrais madame la ministre évoquait une seconde question. La proposition de directive sur le devoir de vigilance des grandes entreprises le Conseil vient d'approuver le 1er décembre dernier une position commune considérablement appauvri visiblement en raison notamment des pressions de la France alors que celles ça c'est 16% des entreprises européennes pratique volontairement une forme ou l'autre de surveillance de l'ensemble de leur chaîne de valeur afin de prévenir les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et l'environnement. Le projet de directive européenne portait l'ambition, de rendre ce devoir de vigilance obligatoire dans toute l'Union. On parlait de 0 abus. Le texte adopté a été largement affaibli la notion de chaîne de valeur a été remplacée par la notion de chaînes d'activités qui n'est pas définie en droit, ce qui ne permet plus d'intégrer les filiales et sous-traitants et fournisseurs aux obligations du devoir de vigilance, le chant du devoir de vigilance nunc Linux l'usage qui est fait des produits commercialisés par les entreprises, ni les activités des clients des entreprises de service, ni les exportations d'armes ou de matériel de surveillance. La référence au secteur financier dans la définition de la chaîne d'activité a été également amoindrie, la liste des services financiers, soumis au devoir de vigilance sera laissé au choix des États. Ainsi, comme le souligne différentes ONG, je cite, de nombreux services financiers seront exclus comme les activités d'investissement ou les activités des partenaires commerciaux des entreprises bénéficiant du service financier. Exemple, tant les banques de leurs obligations de vigilance concernant les activités des sous-traitance des entreprises qu'elle finance alors que par exemple dans le secteur textile ou pétroliers l'essentiel des vols à des violations survient en en lien avec la sous-traitance vous avez Madame la Ministre démenti par voie de communiqué avoir milité pour la sortie des banques du Champ de la directive. Dont acte. Mais comment alors on est on arrivé là que s'est-il passé. Quelle a été et qu'sera Madame la Ministre la position française sur le devoir de vigilance.-- Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre. Monsieur le président de la commission des Affaires européennes. Mes chers collègues. Étape cruciale dans les sanctions affluent infligées à la Russie par l'Occident depuis hier plus aucun navire ne pourra décharger du pétrole russe dans les ports de l'Union européenne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Japon ou de l'Australie. Au terme de difficiles négociations notamment avec la Hongrie, pays de l'Union particulièrement enclavé et qui fait face à de grandes difficultés pour diversifier ses approvisionnements approvisionnement. Un compromis a finalement été trouvé. Seul le pétrole arrivant bah par bateau est concernée par l'embargo. À cet embargo s'ajoute une nouvelle disposition décidée vendredi dernier par l'Union européenne. Les États membres se sont mis d'accord pour plafonner le prix du baril russe à 60 dollars. Ce plafond a été durci avec l'ajout d'une disposition prévoyant de le maintenir. De me, de maintenir 5% en dessous du prix du marché du brut russe. À ce stade s'il le faut nous féliciter de cette décision commune sur un sujet aussi stratégique. Les pays de l'Union faisant face à des situations très disparates en matière d'approvisionnement énergétique et impossibilité de diversification. Nous pouvons également nous interroger sur l'efficacité du dispositif, le baril russe ce négociant aujourd'hui aux alentours de 65 dollars. Plusieurs pays ont d'ores et déjà fait part de leur déception. Autre source d'énergie. La présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne a suggéré aux États de procéder à des ajustements, des conditions d'actualisation du plafonnement des prix du gaz jeudi 1er décembre dans un 1er projet de compromis relatifs au mécanisme de correction du marché. Présenté le 22 novembre à la proposition législative de la Commission européenne prévoit la mise en place automatique d'un plafond sur le prix du gaz, négocier sur le marché des instruments dérivés ITTF lorsque 2 conditions sont réunies de manière simultanée, premièrement le prix de règlement pour les instruments dérivés TTF dépasse 275 euros pendant deux semaines consécutives. Deuxièmement, l'indice TTF hurle PN gaz spot est supérieur de 58 euros au prix de référence du gaz naturel des keffieh au cours des 10 derniers jours précédant la fin de la période de deux semaines sus-mentionnés. Alors que les États membres partisans d'un plafond jugé ces conditions bien trop exigeante. La proposition de la Commission va trop loin pour les pays opposés à tout plafonnement comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Afin de trouver un compromis Prague suggère d'abaisser de 275 à 264 euros. La limite de prix au-delà de laquelle le plafond serait déclenché et de faire passer à 5 jours les deux périodes requises pour activer le mécanisme. Le projet de compromis modifie également le Champ d'application du mécanisme et ne serait ainsi plus limité aux dérider dérivés TTF à un mois mais concernerait également ceux dont l'échéance est compromise entre un mois et trois mois. Enfin, Prague propose de supprimer l'obligation pour les États membres de motifs de notifier à la Commission européenne. Les mesures prises pour réduire la consommation de gaz et d'électricité en cas d'activation du mécanisme. Quelle sera la position de la France sur cette proposition, madame la Ministre. Alors que l'Union européenne entame l'hiver et que certains pays. Et que certains des pays membres font face à des températures allant jusqu'à moins 10 degrés. Les décisions doivent être prises rapidement. À l'instar de la Covid-19. La guerre en Ukraine est un accélérateur des tendances qui structure l'Union européenne. Depuis des mois, la guerre est à nos portes et nous oblige à trouver des réponses adaptées. La démarche engagée par la PFUE lors du 1er trimestre 2022 doit se poursuivre afin de construire une Europe plus souveraine en matière d'énergie, mais aussi plus forte et capable d'agir en matière de sécurité et de défense. À ce titre, nous nous félicitons de l'approbation par la commission d'un investissement de près de 1,2 milliards d'euros dans la recherche et le développement en matière de capacités de défense. 61 projets collaboratifs seront soutenues et bénéficieront de financements du Fonds européen de la défense. Ces projets collaboratifs sont nécessaires pour renforcer à la fois nos fondations industrielle et technologique de défense et leur politique de sécurité et de défense commune. Nous saluons également l'accord trouvé entre les industriels allemands et français sur la face B hein de l'avion du futur SCAF. C'est une excellente nouvelle pour la France mais aussi pour l'Europe de la défense qui a tout de même du mal à prendre son envol. C'est une percée majeure pour l'industrie de la défense de l'Union qui se situe au coeur de la souveraineté européenne souhaitée par la France. Si les blocages de la première phase du projet sont levées il faudra à nouveau négocier pour les phases suivantes du projet et nous appelons de nos voeux des négociations plus apaisée. Pour les prochaines phases. Je vous remercie.--

Madame la présidente Madame la Ministre, Monsieur le Président des Affaires européennes. Mes chers collègues. L'Europe est actuellement plongé dans une crise énergétique inédite. La production des entreprises et menacé et freine la réalisation de l'objectif de réindustrialisation de l'Europe. Les collectivités sont au bord du gouffre et avec elle les services publics Fournier à nos concitoyens qui eux-mêmes seront impactés Tôt ou tard. Puisqu'ils devront bien un jour payer le prix du bouclier tarifaire mises en place pour limiter en urgence l'impact de la hausse des prix. La guerre en Ukraine et tentatives de désorganisation du marché du. De l'énergie par la Russie. Les sanctions prises par l'Union européenne contre le gaz russe ont mis en lumière les mauvaises décisions prises par notre pays en matière de nucléaire, ainsi que les lacunes du Marché commun de l'énergie, en particulier en ce qui concerne le calcul du prix de l'électricité. En effet, alors que le prix du gaz, cette envolée du fait du contexte international. Le coût de l'électricité atteint lui aussi mécaniquement des niveaux jamais vus par le passé, puisqu'il est calculé en fonction du coût de la dernière unité de production qui est généralement une centrale thermique au gaz. La politique des petits pas ne suffira pas pour remédier à cette situation et traiter les conséquences de la crise énergétique sans accepter d'en voir les causes ne ne conduira qu'à une impasse et ne fera qu'aggraver l'état de nos finances publiques. Le marché européen de l'électricité doit donc être réformé urgemment et en profondeur on les décorer des prix du gaz hein dans le but d'éviter que cette crise ne se poursuivent ou qu'elle se reproduise à l'avenir. Pourtant, la Commission européenne n'a à ce jour toujours pas présenté de propositions de réforme et ne devrait pas le faire avant mars 2023, alors que la période hivernale hein sera la plus risquée en terme d'augmentation des prix. Réalisons bien que nous serons cet hiver, confrontés à des risques de Blackout. Et que des délestages seront très certainement mises en oeuvre pour les éviter. C'est du jamais vu, même si le président de la République a tenté de nous rassurer en parle aux des scénarios de la peur. Je comprends bien que le sujet est très sensible parmi les États membres qui ont chacun des mix énergétique et donc des intérêts différents, mais la crise sanitaire nous a prouvé que l'union était capable d'agir beaucoup plus rapidement qu'elle ne le fait actuellement et d'inadaptation du marché est connue de longue date. Il faut accélérer de toute urgence ce volet et la France va engager tout son poids en vue d'aboutir à une solution rapide hein. Je souhaiterais donc savoir Madame la Ministre ainsi une accélération peut être attendu ou si nous devons nous résigner attendent la fin du 1er trimestres 2023 et donc accepter les risques afférents à l'absence d'application d'une réforme durant l'hiver. En outre, pourriez-vous m'indiquer si des pistes commence. Au moins se démarquer, qui est par exemple l'avis du gouvernement sur le système grec qui consisterait à faire reposer négociation du prix sur 2 compartiments de centrales avec d'un côté les centrales à forte proportion de coûts fixes, c'est-à-dire le renouvelable et nucléaire dont le prix de vente serait fixé sur la base d'un appel d'offres en fondée sur le coût moyen de production et de l'autre côté les autres centrales fonctionnant aux énergies fossiles qui aurait un coût variable le prix final l'électricité étant alors formé par une moyenne pondérée des deux. Autrement privilégiant auriez-vous plutôt d'autres prises et si oui lesquelles. Je voudrais en août vous interroger sur une première étape intermédiaire qui pourrait être franchie en cas d'accord sur le principe d'un plafonnement temporaire du prix du gaz du système ibérique. bien évidemment pas d'une réforme structurelle et ce plafonnement n'a vocation à intervenir que dans des cas exceptionnels de très forte hausse des prix. Il aurait néanmoins le mérite d'éviter les situations les plus catastrophiques cependant des désaccords importants persistent entre les États membres, ce qui pourrait encore en retarder l'adoption. En effet, certains pays dont la France est parti. Estime que le plafond fixé pour le moins de 75 euros du MWh est trop haut et que les conditions soient trop difficile à atteindre. L'Allemagne et les Pays-Bas. On en a parlé, ils sont de leur côté plutôt opposés, craignant une hausse de la consommation de gaz et un manque de compétitivité face aux marchés asiatiques et américains qui pourrait entraîner une rupture de l'approvisionnement du continent. Or, le plafonnement du prix du gaz serait justement accompagnée d'un accord de solidarité entre les États membres pour la fourniture d'énergie d'un accord pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et d'un objectif de réduction de la consommation de 15%, ce qui permettrait d'éviter les écueils soulevés par les sceptiques. Par ailleurs, rien n'empêchera en parallèle d'augmenter les livraisons de gaz par le biais de sources dignes de confiance, telles que la Norvège ou l'Algérie. De ce fait Madame la Ministre de Muray-vous optimiste sur l'obtention d'un accord. Les discussions ont-elles avancer et pouvons-nous espérer un assouplissement des conditions et ou un abaissement du plafond ou au contraire est-ce que nous devons nous contenter du mécanisme très restrictif, qui avait été présenté le 24 novembre, au ministre de l'énergie et qui laisse peu d'espoir d'amélioration. Quant au prix du gaz hein. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Gisèle Jourda pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour sept minutes.

Madame la présidente. Monsieur le président de la commission des Affaires européennes. Madame la Ministre, mes chers collègues. Ici dans cette du Sénat. Si on avait dit il y a quelques années lorsque nous avions porté le dossier de proposition de résolution européenne visant à créer le fonds européen de défense. Les réactions de la part. De personnes auditionnées 13 émérite d'anciennes même Ministre des Affaires étrangères avait dit ah mais non. Un fonds de défense parler de défense mais la paix et durable. Malheureusement et je ne reprendrai pas ce qui a été dit. Par mes précédents collègues ben la porte la Si proche de nous, qu'est la nécessité de la réactivité et qu'elle a, donc après le défi sanitaire que l'Europe avait dû faire face nous avons dû donc tenter d'apporter des réponses. Et pas si simple que ça parce que la réactivité européenne, elle est faite de diversité et nous n'avons pas du tout les mêmes objectifs pour certains en tout cas on n'y arrive pas de la même manière et ce n'est pas si évident donc pour moi ce soir je traiterai. Bien entendu, des questions de voisinage, de sécurité et de défense.-- Alors que la défense européenne, n'était plus qu'fantasme pour certains, peu nombreux, qui osaient penser plus loin que l'OTAN et que le Fonds européen de défense que nous nous étions battus pour créé et abondé avait été siphonnés pour faire face au Covid-19, l'Europe hésite enfin décidé à faire siennes les mots d'autonomie et de boussole stratégique.-- Au delà de la de militaires inédite apportée. Aux forces armées ukrainiennes de la décision de faire entrer l'Ukraine et la Moldavie dans le processus d'élargissement. Le 1er semestre a été marquée par l'adoption du 1er livre blanc de la défense européenne cette boussole stratégique européenne a fait l'objet d'un accord unanime des États membres à l'occasion du Conseil européen du 27 mars dernier et il convient de le saluer mais de rester vigilant, je vous renvoie à des statistiques il critique émanant de l'Agence européenne de défense et qui disent que, en terme d'acquisition de matériels on atteint seulement 18% des dépenses de défense. C'est 2 fois moins que l'objectif de 35% fixé par la boussole.-- Ce soutien politique était inédit et doit reposer sur un triptyque, la stratégie, la technique et la crédibilité. L'UE devait prochainement et enfin se doter de la base industrielle et technologique de défense autonome qui sera le fondement technique de son indépendance désormais l'Union doit mettre en oeuvre la feuille de route fixée par la boussole stratégique, c'est une condition nécessaire pour garantir la crédibilité de l'Union sur la scène internationale. la lecture partagée des menaces auxquelles l'Europe doit faire face de le renforcement de la capacité d'action rapide de commandement et de contrôle trois le renforcement de la coopération face aux menaces hybrides dans des domaines tels que le renseignement le cyber l'espace où la lutte contre la désinformation IV la question des investissements qu'meurt en matière de capacités militaires cinq les partenariats stratégiques de l'Union. Il reste une série de questions. Pas très bien abordés et que je résumerai à une phrase. La défense européenne doit-elle être considérée comme un projet visant la coopération ou visant l'intégration. Tant que nous ne clarifie rompe pas ce que notre politique de défense commune est censée représenter au sein de la construction européenne. Nous ne serons pas en mesure de comprendre ce que l'Union doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire ni de départager les attributions respectives de l'Union et de l'OTAN. Parce que le retour de la guerre n'est plus une hypothèse d'école. L'agression inqualifiable rue ceux perpétrés en Ukraine, a dit une preuve sanglante notre action ne sera crédible qu'à condition que nous fassions les efforts techniques et stratégiques nécessaires. Depuis le 23 juin dernier, la politique de voisinage et d'élargissement de l'Union européenne est entrée dans une phase complètement inédite. Se pose alors la question suivante qu'mal valorisé dans le processus d'élargissement. Les efforts incontestables réalisés par l'Ukraine et la Moldavie, dans le cadre du Partenariat oriental. Est-ce qu'on prend en compte les acquis obtenus ou est-ce qu'il reparte à 0 dans cette presse procédure procédure longue alors que dans l'accord d'association, ils avaient déjà rempli certaines crises critères. Bon élève du Partenariat oriental, quid de la Géorgie pourquoi et nous disons pas qu'elle ne remplissait pas les critères. Ce serait inexact. Depuis octobre, était organisée la première réunion de la communauté politique européenne voulue par le président Macron permettant selon lui aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle socle de valeurs de trouver un nouvel espace de coopération politique de sécurité de coopération.-- Prompt à saluer toute initiative de coopération. Je m'interroge sincèrement Madame le Ministre sur le fonctionnement de nos instances européennes et internationales existantes ne sont-elles pas, c'est déjà être cet espace de même périmètre que le Conseil de l'Europe ne s'agit-il pas d'un doublon comment seront vécu les futures réunions prévues en Moldavie et en Espagne. Je m'interroge, si nous n'a n'y arrivons pas à trouver des positions communes à 27. Allons nous y arriver à 44. Puis il y a un risque grave, celui que l'Union ne s'écartèle sous le poids des ensembles régionaux devenus trop puissant ou qu'elle ne se détruisent, en raison d'intrusion de superpuissance bien mieux organisé que nous. Le succès de la nouvelle phase de la politique d'élargissement qui s'est ouverte cet été reposera sur la capacité de l'UE à faire preuve de pragmatisme et à développer des coopérations concrètes avait nos partenaires la CPE peut en être l'un des éléments entre une adhésion accélérée illusoire et une procédure interminables aux effets délétères. La communauté politique européenne à au moins le mérite d'Harry. Mais rapidement l'UE et les pays aspirant à la rejoindre. Je finirai. En demandant un plan de relance pour le partenariat oriental, puisqu'il y avait un accord d'association en train d'être donc établi avec l'Azerbaïdjan ou à des. N'. Non pas le par 9 tenariat orientale s'étonne Toniutti ne le négligeons pas. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean Michel Arnaud pour le groupe Union centriste pour 7 minutes.-- Madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues.-- À quelques jours du Conseil européen. Nous tenons ce traditionnel débat parlementaire visant à éclaircir les différents points qui seront abordés. Pour commencer. Le conflit russo-ukrainien demeure le plus grand défi actuel de l'Union européenne. Dans une guerre unilatéralement déclarée par la Fédération de Russie. Nous devons évidemment rester aux côtés du peuple ukrainien et de son gouvernement. Alors que les soldats des 2 armées creusent des tranchées et les combats font rage comme à Bakhmout où opère la sinistre milice Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine une issue diplomatique semble impossible à court terme. Nous y sommes donc. La guerre de mouvement fait place à une guerre de position. Ces termes ne sont pas anodins pour nous Français, puisqu'il renvoie au 1er conflit mondial qui a marqué à jamais notre pays. Notre rôle aujourd'hui est de puiser dans les leçons du passé pour mieux préparer l'avenir. Il s'agit de prévenir tout embrasement militaire à l'échelle continentale. C'est pourquoi le soutien tant militaire qu'humanitaire en faveur de l'Ukraine doit se poursuivre s'intensifier. Aussi pour parapher paraphraser la devise européenne. Nous avons l'impérieuse nécessité de rester unis dans la diversité. Unis comme ce fut le cas lors de l'adoption de plusieurs paquets de sanctions dont les effets limités reste perceptible puisque le PIB russe a diminué de 4% en 2022. Solidaire aussi en matière de défense, l'envoi de troupes françaises. Italienne ou encore belge dans les États minime trompe de la Russie participe à maintenir une posture face commune face à Moscou. J'ai à cet instant une pensée particulière pour nos soldats français mobilisés et tout particulièrement pour le 4ème régiment de chasseurs alpins de Gap, dans mon département des Hautes-Alpes qui stationnent actuellement en Roumanie. Mes chers collègues. Quand les démons du passé frappent aux portes du présent. Il est de notre devoir de démocrates de faire triompher la raison sur la passion l'humanité sur la brutalité. Oui, cette guerre a définitivement été un révélateur des forces et faiblesses de l'Union européenne à tout niveau. Si j'ai mis en avant la réaction unanime et concertée des États membres. Face à cette agression russe. Il ne faut pas pour autant occulter nos erreurs collectives et nous devons tirer les enseignements. Je pense par exemple aux décennies le débat autour de l'autonomie militaire de l'Union qui nous font aujourd'hui défaut. Si la France a toujours été pro-actif sur ces sujets. Nombres d'États membres a souvent repoussé les discussions aux calendes grecques l'accroissement des dépenses militaires annoncées par l'Allemagne ou encore la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande vont dans le bon sens mais ce n'est que le début d'un processus. Autonomie stratégique au niveau européen également une assurance vie face au au futur mutation Jo pour logique géopolitique pardon dans un ordre mondial toujours plus troublé néanmoins autonomie ne signifie pas isolationnisme. C'est pourquoi je m'inscris dans les récents propos du président de la République Emmanuel Macron qui, à l'occasion de sa visite d'État aux États-Unis a appelé rend à renforcer l'intimité stratégique entre les 2 côtés de l'Atlantique. Nous sommes, a-t-il dit. Et je suis d'accord avec lui des frères d'armes. La nécessité de construction d'une autonomie s'applique également au secteur énergétique comme ça été évoquée par un certain nombre de collègues précédemment. Le développement des énergies renouvelables au sein d'un mix énergique énergétique doit être favorisé à l'échelle européenne. En effet les situations s'avère très disparate. Alors que les besoins de gaz hongrois dépasse à 80% dépendent à 80% du gaz russe. D'autres États tels que la France possède une autonomie énergétique relative, je dis bien relative car il n'est pas uniquement question de production mais de l'ensemble de la filière des matières premières à la commercialisation, en passant également. Il moment par le traitement des déchets nucléaires. Car oui, vous l'avez sans doute vu dans la presse récemment. L'unique entreprise capable de recycler l'uranium de nos centrales nucléaires et russe. Le groupe Orano continue donc d'expédier de l'uranium vers l'usine de Seversk en Sibérie appartenant au groupe Rosatom. En parlant de dépendance économique. Je souhaite également évoquer la récente annonce du gouvernement américain portant sur l'inflation réduction Act. Ce plan de réformes qui vont aussi qui couvre aussi bien la santé que le soutien aux entreprises prend tout particulièrement un volet climat. Près de 400 milliards de dollars serviront à financer des mesures sur 10 ans, qui doivent permettre aux États-Unis d'atteindre leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les particuliers, cela signifie par exemple une aide de 7500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique ou un dispositif de soutien à l'installation de panneaux solaires. Jusqu'ici tout va bien. Mais ces mesures ne concernent pas uniquement les produits et services provenant du sol américain ou nord-américain. Cette véritables clause de préférence nationale n'est pas sans conséquences pour les Européens. Parce qu'elle met en danger les industriels. L'administration Biden va favoriser les classes américaine par rapport aux BMW allemande ou Renault ou Peugeot française il y a surtout un risque de délocalisation massive d'entreprises européennes ou américaines ayant investi en Europe et qui préféreront fabriqués sur le sol américain, pour pouvoir bénéficier de ces aides. Ces mesures ouvertement protectionnistes vont et ça a été à plusieurs reprises, rappelé à l'encontre des principes de libre-échange de l'OMC. C'est du moins ce qu'ont déclaré également les ministres de l'économie allemand et français. Face à cet état de fait nous européens devons réagir soit en négociant des dérogations comme ça a été le cas pour les Canadiens ou les mexicains ou bien ce qui a été proposé par le président de la République. Nous devons établir des dispositifs similaires afin de sauvegarder les industries européennes et affirmé la la place du Vieux Continent dans la compétition mondiale face à la Chine. J'attends effectivement Madame la Ministre des précisions à cet effet. Là dans le dernier dossier que je souhaite aborder devant vous n'est pas forcément le plus médiatisé, mais c'est celui qui a le plus d'écho dans les territoires ruraux. La nouvelle politique agricole commune pillé la construction européenne, l'ambition de l'auto-suffisance alimentaire a toujours animé cette dernière bien que plus de 387 milliards d'euros, il soit consacrée jusqu'en 2027 avec des objectifs sociaux et environnementaux ambitieux 2 écueils et non des moindres persiste. Les nouveaux objectifs s'inscrivent dans le Pacte Vert européen visant à favoriser la transition écologique. Dans cette optique, une étude du jogging sweat-shirt Center conclut que la mise en place de cette démarche entraînerait une réduction de la production de 10 à 15% dans les filières céréales, oléagineux viande bovine produits laitiers de plus de 15% dans le porc et la volaille. Et de plus de 5% dans les légumes et cultures permanente. J'ai l'air dans dans la ministre la transition écologique dans le domaine agricole n'est pas de produire moins mais de produire mieux, où il faudra bien nourrir nos citoyens et si nos agriculteurs produisent moins au non la réduction des et des émissions de gaz à effet de serre, nous aurons recours aux importations depuis l'étranger dont l'empreinte écologique est bien supérieur, l'écologie doit certains toutes nos politiques agricoles et elle doit se conjuguer aussi avec les défis alimentaires à venir. à la différence de l'ancienne Pâques la nouvelle prévoit que ce sont les États qui définit les priorités du pays et les critères sur lesquels seront versées les aides vertes dans le cadre d'un plan stratégique national. Que les États étaient une marge d'appréciation d'adaptation pour la bonne application de la plaque, c'est une chose mais le fait que chaque État fixe sa feuille de route en est une autre. Concrètement, nous assistons à une renationalisation de cette politique qui n'a de, de quand même plus que les, enfin j'en appelle donc le gouvernement afin qu'il engage tous les moyens possibles pour préserver notre culture et nos agriculteurs je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur André Reichardt. Pour le groupe Les Républicains et pour cinq minutes. C'est le président Madame la Ministre, mes chers collègues. Les discussions du prochain conseil européen sur une nouvelle fois dominée par la guerre en Ukraine et ses conséquences sur notre continent. Néanmoins, les chefs d'État et de gouvernement débattront aussi à cette occasion des relations qu'entretient l'Union avec son voisinage méridionale. Nos Liens avec la rive sud de la Méditerranée et au-delà avec le continent africain revêtent naturellement de multiples dimensions. l'actualité récente, celle du fiasco. Ce qu'il faut bien appeler le fiasco de l'Océan Viking mais aussi celle, un peu plus anciennes du drame de Melilla en juin dernier, vient nous rappeler à quel point la question migratoire reste prégnante. 7 ans après le déclenchement de la crise de 2015. Nous, nous ne pouvons que constater combien l'Europe reste englué dans des contradictions, incapable d'opposer une réponse commune à 10 mouvements migratoires qui semble toujours plus. Dès 2016, pourtant un 1er paquet de réformes avaient été proposé par la Commission Juncker mais malgré un certain nombre d'accord. Entre le Parlement et le Conseil il s'est finale il s'est au final heurté au mur des dissensions concernant la prise en charge des demandeurs d'asile. La Commission von der Leyen a donc repris le flambeau, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ces propositions sont elles aussi bloquées depuis 2 ans. La présidence tchèque Czech comme avant. Comme avant elle, la présidence française ne ménage pas ses efforts pour pas parvenir à un compromis quelques progrès sont certes heures salué comme par exemple sur Eurodac ou sur les règles le règlement filtrage mais l'équilibre global. Indispensable pour que la réforme puisse aboutir semble toujours largement hors de portée. Équilibré entre États. Bien sûr, mais aussi entre institutions car le Conseil malgré ses divisions sur l'aspect solidarité se retrouve largement sur certains points fondamentaux comme la protection des frontières extérieures, le renforcement de la politique de retour ou l'attention accrue portée au modus operandi de certaines ONG de Méditerranée qui s'avère parfois je dirais même, souvent contraires aux règles et procédures définies par les conventions internationales. Cette approche est malheureusement loin d'être par. Au Parlement européen, voire même au sein de la commission ou prévoit une ligne différente qui s'apparentent parfois une consécration de facto d'un nouveau droit à la migration. Je dis bien droit à la migration. Elle semble rejeter par principe un postulat pourtant fondamental qui est que nul ne doit pouvoir entrer ou s'installer sur le sol européen sans y avoir été au préalable légalement autorisé entre ces 2 conceptions divergentes. L'Europe semble toujours incapable de trancher. L'agence Frontex et en particulier son désormais ex-directeur exécutif ont fait les frais de cette opposition entre le Conseil, la Commission et le Parlement Font les frais aussi de ces injonctions politiques contradictoires qui n'ont cessé d'en découler alors même que cette même agence Frontex comptabilise vous le savez, sur une année 281.000 passages illégaux des frontières de l'Union en progression, excusez du peu de 77% sur l'année précédente. Cette ambiguïté. Clairement ambiguïté de l'Union maintient notre continent dans un tragique état de fragilité face au phénomène migratoire et le condamne à un certain nombres de psychodrame. La récente crise franco-italienne en est une parfaite illustration et contraint malheureusement à rechercher à rechercher de vagues solution d'attente. La commission a ainsi présenté le 21 novembre dernier un plan d'urgence en 20. Censé répondre à la hausse des flux en Méditerranée au mésentente des États, concernant les opérations de recherche et de sauvetage, un plan qui dans les faits, ne propose rien de véritablement concret ni de très nouveau, notamment par rapport aux mécanismes volontaires de solidarité mis en place en juin dernier. En attendant, le nombre des arrivées des demandes d'asile explose à nouveau. Quant à la politique de retour, la présidente je check constate malheureusement que malgré les outils mis en place ces résultats restent médiocres Madame la Ministre les institutions européennes ont signé une feuille de route avec en point de mire un accord d'ici février 2024 soit l'ultime limite avant les prochaines élections européennes. Ce calendrier avant tout basé sur des considérations politiques bien sûr a toutes les chances malheureusement de ne pas être tenu. Il y a pourtant urgence à conclure ce dossier qui n'a que trop duré et qui sape chaque jour un peu plus la crédibilité du projet européen vis-à-vis de nos concitoyens. N'oublions pas non plus qu'avec la crise de 2015, ce sont les fondations mêmes de l'espace Schengen qui ont vacillé menaçant d'emporter avec elle. Le principe de libre circulation. La question de l'asile et d'immigration reste donc indispensable de celle du fonctionnement de l'espace Schengen, la réforme engagée, bien que loin de la remise à plat voulu il y a quelques mois par le président de la République apparaît néanmoins utiles mais elle aussi n'avance que lentement. Et alors qu'elle n'a pas encore mais était mené à bien la Commission et le Parlement européen viennent de donner leur aval à l'adhésion de la Croatie son en fait collègue tout en préconisant également l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. Selon toute vraisemblance le Conseil se prononcera, dans deux jours sur cette question, madame la Ministre, quelle sera la position défendue par la France à cet égard, je vous remercie.-- Merci cher collègue. Et la parole est maintenant à la présidente. Pascale Gruny. Pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, hein. Monsieur le président de la commission des Affaires européennes, chers collègues. Les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles dans un contexte géopolitique et économique toujours très Si la guerre en Ukraine sera une nouvelle fois au menu des échanges avec l'entrée en vigueur du dernier train de sanctions à l'encontre de la Russie, les échanges porteront aussi sur les tensions commerciales entre Européens et Américains. En se rendant aux États-Unis. Emmanuel Macron espérer convaincre Joe Biden de renoncer à son inflation réduction Act. Mais il n'a pu que constater une nouvelle fois la posture hyper-protectionniste des Américains dont il avait déjà fait l'amère expérience en 2021 lors de l'annulation du contrat du siècle avec l'Australie. Les priorités de Joe Biden ont toujours été claires, d'abord la politique intérieure, ensuite la chute. La Chine est loin derrière éventuellement l'Europe cette posture des Américains renvoie l'Europe à ses propres faiblesses et à l'impérieuse nécessité pour elle de réagir si elle ne veut pas finir par devenir invisible invisible sur la scène internationale. Face à l'ampleur des plans américains de nature protectionniste. Aggravée par un choc négatif de compétitivité des prix de l'énergie, l'Europe doit soutenir puissamment son industrie et appliquée, elle aussi une préférence pour les productions localisée sur notre continent. Encore faudra-t-il que l'Europe puisse lever des moyens comparables à ceux des États-Unis, quand nous autorisons un financement public de 5 milliards d'euros pour l'hydrogène Vert, Washington met 100 milliards de dollars sur la table, le chemin semble donc encore bien long. Puisqu'il est ici question de souveraineté industrielle. Je voudrais vous interroger sur 2 sujets importants qui ont fait l'objet de travaux récents au Sénat, la santé et le numérique. En matière de santé, notre pays fait actuellement face à des ruptures d'approvisionnement concernant de nombreux médicaments et c'est le cas notamment de la cortisone et des antibiotiques, alors que la situation est similaire chez nos voisins. La Commission européenne tarde à proposer une révision de la législation pharmaceutique et un plan d'action à l'échelle de l'Union pour lutter contre ces pénuries qui passe par une plus grande maîtrise des approvisionnements et de la production. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est aujourd'hui, ce que peut faire la France pour inciter la Commission à prendre davantage en compte ce problème. Par ailleurs, la Commission a présenté une proposition de règlement visant à établir un espace européen des données de santé. Le Sénat et je serai avec ma collègue Laurence Harribey entend se saisir de ce sujet pour garantir la. Protection des données à caractère personnel. En effet si nous comprenons bien l'enjeu que représente l'utilisation de ces données pour favoriser la recherche médicale. Il est tout aussi indispensable d'en préserver la confidentialité pour assurer la protection des libertés individuelles. Les cyber attaques récurrentes menée contre notre système de santé. La dernière en date vise l'hôpital de Versailles depuis samedi démontrent que le sujet doit être pris très au sérieux. Nous devons nous contre c'est à coeur sans scrupules qui n'hésitent plus à diffuser sur le dark Net des données confidentielles concernant les patients. Pouvez-vous nous dire quelle est la position que défend actuellement le gouvernement français dans le cadre des négociations au Conseil sur ce texte et notamment ce qui concerne l'hébergement des données. En matière de numérique. La Commission européenne a également présenté une proposition de règlement visant à améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Ces plateformes numériques modifie la relation salariés-employeurs classique et ont donc un impact important sur notre législation, notre vigilance est nécessaire pour garantir la protection des travailleurs. Pouvez-vous nous donner des informations concernant l'évolution des négociations sur ce texte. Ça intéressera aussi ma collègue Laurence. Aujourd'hui l'Union européenne, tout comme les États sont confrontés au défi que représente l'utilisation accrue des technologies du numérique développé le plus souvent par des opérateurs étrangers. On le voit aussi bien sur la question des travailleurs de plateformes que sur l'espace européen des données de santé. La question de la sécurité qui est à l'ordre du jour du prochain conseil européen ne peut être dissociée de la question de la souveraineté européenne tant sur le plan sanitaire que sur le plan numérique. Cette question doit désormais devenir central dans toutes les discussions. Nous comptons sur le gouvernement français pour éveiller de près. Merci de votre attention.

Je ne savais pas si je devais dire madame la présidente, monsieur le président. Donc ce sera madame la présidente. Madame la Ministre. Monsieur le Président rap Chers collègues. Le Conseil européen des 15 et 16 décembre va être largement consacré aux questions de politique étrangère de sécurité et de défense. évidemment, la guerre en Ukraine et les relations. Que l'union de l'Union pardon avec les pays de son voisinage méridional. Il est cependant prévu que les chefs d'État et de gouvernement aborde également certaines questions économiques concernant l'énergie. À l'évidence, toutes ces questions sont liées entre elles et plus lourde et urgente les unes que les autres. Nos concitoyens attendent surtout des dirigeants européens, qu'il fasse preuve de fermeté dans la défense des intérêts de l'Union et d'efficacité dans la prise de décision.-- La solidarité avec le peuple ukrainien doit être sans cesse réaffirmée. Qu'on le veuille ou non tout signe contraire témoignant d'un début de lassitude de nos opinions publiques ou d'une certaine. Irrésolution de l'Union serait perçu par les Russes, comme un signe de faiblesse.-- Nous n'avons donc pas d'autre choix que de poursuivre dans cette voie. Et de maintenir à tout prix l'unité du bloc tant qu'une issue satisfaisante. N'aura pas été trouvées dans des termes acceptables pour l'Ukraine.-- Le président de la République a récemment répété qu'il entendait maintenir un dialogue Direct. Avec le dirigeant russe. Je veux croire qu'il le fera avec le soutien explicite de ses partenaires européens. Et des autres alliés de l'Ukraine. L'exercice est délicat car il faut éviter d'ajouter de la confusion à la confusion. Les postures narcissique et la volonté de se donner une importance personnel. Ne doivent tenir aucune place dans ce genre d'exercice. Le Conseil européen de décembre sera l'occasion pour le chef de l'État, le chef d'État et de gouvernement. D'envisager un paquet supplémentaire de sanctions. Le 9ème contre la Russie. Toute sanction, quelle qu'en soit la nature et l'ampleur soulèvent cependant 2 questions essentielles. Celle de de son efficacité pour amener le pays. Qui en est la la cible. À résipiscence et celle de ses éventuelles répercussions négatives sur les pays qui adopte les sanctions eux-mêmes.-- Il me semble que sur l'un et l'autre point, la pertinence dès huit paquets de sanctions adoptées jusqu'ici par l'Union n'a pas encore été totalement démontré. Loin s'en faut. Il serait bon que l'examen d'un nouveau paquet d'éventuelles sanctions fournissent l'occasion d'un bilan réaliste.-- La question vitale de l'énergie et bien sûr lié aux développements géopolitiques récents mais elle ne s'y résume pas. Le tarissement de nos approvisionnements en gaz et pétrole de Russie a surtout surtout mis en évidence. Les mauvais choix politiques fait en Europe et en France en particulier au cours de la dernière décennie marquée par un Bordeaux Pro quatre programmée injustifiable de la filière nucléaire. Une aggravation inconsidérés également surtout de la part de l'Allemagne. De la dépendance gazière vis à vis de la Russie. L'explosion des prix de toutes les sources d'énergie que nous subissons actuellement se conjugue à d'autres facteurs pour attiser le foyer d'une inflation galopante qui affecte de plus en plus durement les les entreprises comme les familles. Enrayer ce processus infernal devrait être l'une des premières priorités des dirigeants européens. La solidarité est évidemment de mise, même s'il est apparu récemment que les intérêts des uns et des autres peuvent sérieusement diverger voir se heurter. Nous attendons de ce Conseil européen qu'il propose des solutions forte et cohérente. Susceptibles de manifester rapidement leurs effets sur le marché des produits énergétiques. Par ailleurs, toute discussion entre les chefs d'État et de gouvernement sur les relations de l'Union avec son voisinage méridionale est particulièrement. Avec les pays du Maghreb devra porter en priorité sur le problème de la gestion des flux migratoires. la question de l'accueil des candidats à l'immigration en Europe et de plus en plus urticantes. Elle envenime aussi bien au débat de politique interne. En faisant le jeu des extrêmes des 2 bords que les relations diplomatiques entre les États principalement concernés pas au sein de l'Union. fait que efficacement contre ce phénomène et contre les réseaux criminels qui l'entretiennent la coopération des pays d'origine. Être indispensable. Elle n'est cependant pas à la hauteur de ce que l'Union serait en droit d'attendre. Le refus de réadmission, le plus souvent manifestée par ces derniers, suite aux décisions d'expulsions prises par les autorités des pays européens sont tout simplement intolérables. Les accords de réadmission et la mise en oeuvre d'une coopération judiciaire et policière étroite. Devrait constituer pour l'Union, une condition sine qua none à l'ouverture commerciale de notre marché intérieur. Aux marchandises de ces pays et des autres mécanismes d'aides européennes à leur développement économique. Ou donc Madame le Ministre quelques-unes des grandes préoccupations que nous souhaiterions voir porté par le président de la République à l'occasion de cette importante réunion du conseil. Parfait, merci. Merci cher collègue. La parole est à madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargé de l'Europe.-- merci madame la présidente. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des Affaires étrangères. Dames les sénatrices messieurs les sénateurs, merci vraiment pour vos interventions et questions. je vais tâcher de répondre en commençant par les points à l'ordre du jour au conseil européen, avant de revenir sur les autres sujets d'actualité sur lesquels vous avez eu la gentillesse de m'interroger. Alors vous avez pour la plupart d'entre vous tout d'abord évoqué la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Je voudrais le redire devant vous, la France continuera de soutenir l'Ukraine. Comme le disait le sénateur Marie d'une façon humaine. J'avais un soutien humanitaire pardon militaire et financier et je crois qu'il faut se rappeler du soutien humanitaire dans les comparaisons parfois trop hâtives. Car l'Europe est le seul continent qui accueille 2 millions de réfugiés. Continueront de la soutenir dans la durée puisque comme. La sénatrice Guillotin et le vice-président Alizard ont souligné. La guerre risque d'être longue et j'aurais dû être. Ajouté. Pour Pour vous répondent monsieur Alizart d'ailleurs que lorsque nous parlons de de soutien de défense. Nous parlons évidemment de préférence européenne, par exemple dans le cadre et dire pas et nous y prêtons une attention toute particulière. Monsieur le Sénateur Cadec hein vous avez mentionné certaines. Paroles sur l'Ukraine. Je je veux le répéter ici la paix se fera dans les conditions de l'Ukraine. Et quand l'Ukraine suédois hein c'est ce qu'a dit le président de la république comme tous nos partenaires.-- Enfin. Comme vous savez, l'Union européenne a décidé et travaille pour soutenir l'Ukraine dans cette guerre avec tous ses alliés avec nos partenaires du G7, avec l'Australie et dans ce cas, nous avons décidé de plafonner les prix du pétrole russe ce plafond a été fixé, vous le rappeliez, monsieur le sénateur Kern à 60 dollars.-- Cette mesure, contribuera à réduire la capacité de la Russie à mener sa guerre en diminuant fortement ses revenus issus du pétrole et je dois dire qu'elle a déjà contribué à faire baisser les prix, monsieur de Montgolfier puisque les prix du brut ont atteint un record. Bah aujourd'hui.-- Pour la suite. L'Union européenne continue de travailler à de nouvelles mesures après déjà 8 paquets. De sanctions qui pèsent sur le régime russe. Il y a plusieurs options supplémentaires à l'étude, notamment la restriction d'exportation dans les domaines technologiques bancaire, des services ainsi que de nouvelles désignation de responsables politiques, militaires et économiques russes qui soutiennent la guerre. Monsieur le président, Alizard, Monsieur le Sénateur, Arnaud, vous l'avez tous les 2 souligné c'est l'affaiblissement de la Russie à moyen terme que nous viserons que nous visons et que nous obtiendrons. Monsieur le Président. Hein vous m'avez interrogé sur la mise en place d'un tribunal spécial pour les crimes d'agression de la Russie.-- La lutte contre l'impunité pour les crimes commis en Ukraine à la suite de l'agression de la Russie et pour la France une priorité. Nous nous sommes mobilisés en soutien, tant de la justice ukrainienne que de la Cour pénale internationale. Et concernant la proposition de créer un tribunal spécial. Nous avons commencé à travailler avec nos partenaires européens et ukrainiens. Vous savez que nous avons reçu l'envoyé spécial à ce sujet ukrainien. Il s'agira. Évidemment, d'obtenir le plus large consensus possible au sein de la communauté internationale. Sur les enjeux énergétiques qui je crois avec vos nombreuses interventions et là je peux regarder tout le monde. Il me semble Comme vous le savez si vraiment au coeur de nos priorités communes et j'ai rappelé les différents textes, sur lesquels les ministres de l'énergie ont travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines. évidemment l'importance de préserver un cadre de concurrence équitable, comme l'ont rappelé les sénateurs mais de vielle et avec de la solidarité comme l'a rappelé de sénateurs faire Nick. Monsieur le président aura pas madame la sénatrice Guillotin, vous avez mentionné le mécanisme de plafonnement du gaz. Il ne va pas assez loin. Nous en sommes d'accord. Il y a certes une réforme de l'indice du gaz pour mieux refléter les prix à la fois du gaz par gazoduc et du GNL. Mais il est clair que ça ne va pas nous allons continuer d'appuyer pour faire baisser les prix du gaz et nous allons. Continuer d'endosser la palette d'outils qui existent déjà et qui vont au déjà contribué à faire baisser les prix. Je pense à la plateforme d'achat conjoint qui bien sûr nous donne un pouvoir de marché important je pense aux discussions avec les partenaires stables comme la Norvège comme les États-Unis. Et puis je pense évidemment à l'accélération du renouvelable qui va accroître notre indépendance. Je crois que le sénateur Marie l'a mentionné en particulier. Monsieur le Président rap hein. Monsieur le président Laurent Monsieur le sénateur va vous m'avez interrogé sur l'état des négociations sur la réforme du marché d'électricité nous sommes d'accord. Cette réforme est absolument essentielle, puisqu'elle va nous permet de découpler durablement les prix de l'électricité des prix des énergies fossiles. Il se trouve que la Commission nous a donné un calendrier précis, assez précis pour cette réforme une consultation va être va être lancée sur la base d'un 1er projet d'ici quelques jours et sur cette base la Commission fera une proposition législative au mois de mars. cela prend un peu de temps puisqu'il y a non seulement consultations mais aussi étude d'impact. Monsieur le sénateur, va. Et à ce propos, je crois que nous nous dirigeons vers quelque chose qui ressemblera aux contrats pour différence.-- En tout état de cause, cette réforme sera adoptée avant les élections européennes au printemps 2024 et elle elle s'appliquera donc pour l'hiver 2024 2025. Il va donc falloir que nous travaillons à une solution pour l'hiver 2023 2024 pour que les prix d'électricité soit maîtrisée. Ça peut être une prolongation des mesures de captation de rente de la ronde des énergéticiens que nous avons adopté cet hiver.-- À ce propos, il est vrai que l'inflation générée par l'énergie nous soucie et aura sûrement des impacts elle on a déjà sur les projets financés par les PNR. À ce stade nous n'avons envisagé que des modifications marginales du cadre financier pluriannuel pour pouvoir préserver nos priorités mais évidemment nous suivrons attentivement. À moyen terme hein. Monsieur le Président. Alizard c'est la transition énergétique effectivement qui nous assurera la sécurité et pour cela l'autonomie la plus grande possible et là, ainsi que la diversification des sources d'énergie. Il n'y aura pas et plusieurs d'entre vous l'ont souligné, pas de retour au Business as Usual.-- Madame la sénatrice Véronique Guillotin, vous m'avez interrogé sur les relations avec la Moldavie. Vous l'avez dit, vous êtes présidente du groupe d'amitié avec ce pays. La Moldavie s'est vu octroyer le statut de pays candidat lors des conseil européen des 23 et 24 juin. Elle a maintenant à mettre en oeuvre les neufs mesures énoncées par la Commission européenne dans son avis du 17 juin sur la demande d'adhésion moldave, qui porte sur la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, la criminalité organisée et l'influence des oligarques. La réforme de l'administration publique, la réforme de la gestion des finances publiques et de la protection des droits de l'homme. J'ai bien conscience que cela paraît beaucoup est important mais c'est important pour préserver l'État de droit à nos frontières et dans l'Union et nous soutiendrons et nous soutenons les efforts de la Moldavie pour mettre en oeuvre ses réformes.-- Madame la sénatrice Jourda, vous m'avez justement interrogé sur l'articulation de la CPE avec les autres organisations notamment le partenariat oriental mais également le Conseil de l'Europe et vous n'avez pas manqué mentionné l'OSCE si mon souvenir est bon mais je le rajoute. La FCPE. N'est pas une organisation multilatérale concurrente de ces organisations.-- Et c'est le souhait très clair d'une majorité de nos partenaires d'ailleurs que de préférer un format très souple qui soit plus proche de celui du G7 ou du G20, qui est comme vous le savez, n'a pas de secrétariat permanent. Nous sommes attentifs à la bonne articulation des travaux et du calendrier de la CPE avec ceux du Conseil de l'Europe. Comme de l'Ouest. C'est comme du Partenariat oriental. Je crois qu'il faut distinguer les objectifs OSCE sécurité conseil état de droit et CPE, il va y avoir à la fois un espace politique notamment pour discuter par exemple des sujets, Arménie, Azerbaïdjan ou des sujets des. des mers dans ses, dans dans cette zone là et s'il a été très utile, vous vous le rappelez. Le 6 octobre pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais également de projets concrets. Notamment on là je le mentionnais tout à l'heure l'éventuelle itinérance graduelle pour ces pays. Mais aussi par exemple des infrastructures. je crois qu'il faut ajouter qu'il y a un grand appétit de beaucoup de ces pays de l'Ukraine de la Moldavie et des Balkans occidentaux pour pour cette communauté politique européenne qui leur permet de bénéficier de notre voisinage. Au fur et à mesure que l'élargissement se fera.--

au moins il y a quelque chose de consensuel. Vous avez mentionné l'une. Réduction Act. Et je crois d'ailleurs certains et on on effectivement dit que cela s'ajoutait au différentiel de compétitivité qui est créée par le choc sur les prix de l'énergie. Il est vrai et j'ai eu vous oublié, madame la présidente Gruny, j'espère que vous me pardonnerez, je viens de m'en rende compte. Je crois qu'il y a plusieurs choses à avoir en tête la première chose c'est effectivement il y a quelques marges de manoeuvre dans l'application de cette loi américaine dans ce qu'elle va être traduite en décret mais ses marges de manoeuvre et je crois que vous en avez parfaitement conscience sont assez faibles. Nous disposons ensuite d'outils européen d'abord les outils Antibes subventions certains d'entre vous se sont inquiétés d'une. Possible guerre commerciale et c'est pour ça que les anti les outils anti-subventions seront manier avec précaution. Vous avez également mentionné le fonds souverain qui avait été mentionné par la présidente de l'Union européenne dans son discours de l'état de l'Union en septembre. La plupart des pays, comme vous le savez peut-être, j'étais au Conseil compétitivité qui en a discuté la semaine dernière sont en faveur non seulement d'augmenter d'abord d'accélérer la mise en place du fonds souverain d'augmenter les investissements dédiés. Plusieurs d'entre vous ont mentionné les montants de Pierre et aussi d'accélérer la délivrance de ces pièces comme du fonds souverain en particulier parce que les États-Unis avec une flèche une réduction Act mettent en place des crédits d'impôt qui sont évidemment beaucoup plus rapide que le montage de projet. Par ailleurs. Comme vous savez ces projets sont aussi beaucoup destiné à la transition. Notamment dans le domaine de l'hydrogène et des batteries. Et à cet égard d'ailleurs, je je dois féliciter le soutien du Parlement européen, notamment lorsqu'il s'est agi, je vire un peu sur la transition de la déforestation. Et et du soutien apporté par le député-. Qu'enfin. Sur la Chine. Monsieur le sénateur Gattolin entre autres je crois. monsieur le président a les armes a posé énormément de questions, il faut le reconnaître. Vous savez que nous avons ce triptyque de coopération de concurrence et de rivalité systémique lors du dernier Conseil européen le président de la République a été extrêmement vocale sur l'augmentation du poids de la rivalité systémique dans notre dans nos relations avec la Chine, ce qui en concret et se traduit effectivement par du travail à renforcer à la fois les clauses miroirs. À la fois les la réglementation sur l'accès à nos marchés publics, et bien évidemment a considérer que dans le futur on pourrait aussi s'intéresser de plus près sur les outils de contrôle d'exportation ou de filtrage d'investissement.-- Les. Un mari et ma de. Interrogé sur le franco-allemand. Je dois dire que la semaine passée était quand même le témoignage d'une. Intense relation franco-allemande puisque la ministre des Affaires étrangères. Est venu à Paris voir la Ministre Colonna. Le ministre des finances et le ministre de l'Économie, sont allés voir le ministre Bruno Lemaire. La Première ministre hein s'est rendu à Berlin et je l'ai accompagnée et c'est vrai qu'il y a un travail intense. Dans la perspective du prochain conseil des ministres franco-allemand, dont la date n'est pas encore fixée, mais nous avons tous en tête qu'il y a aussi une date importante qui est celle des 60 ans. Du traité de l'Élysée et les travaux s'intensifie dans le domaine de la défense du spatial de l'énergie de la culture de l'éducation. et beaucoup d'autres encore dont on pourra parler une autre fois mieux. Plus pareil. Les sénateurs Marie m'a également interrogée sur le pacte de stabilité et croissance nous irons nous retrouvons dans les propositions de la commission les principes auxquels nous sommes attachés, croissance, investissements et soutenabilité. Nous avons un cadre commun avec des trajectoires personnalisée qui vont nous permettre effectivement de mettre en oeuvre les investissements dont nous avons besoin nous ça peut être les investissements de la transition énergétique. Nos amis allemands peut-être plus la défense en plus de la transition énergétique et ce cadre devrait permettre cette souplesse bien sûr, le diable est dans les détails et nous attendons encore quelques détails.-- Voilà pour. Le Conseil européen. Je vais passer aux questions plus particulières et notamment monsieur le président, Pierre Laurent et Monsieur le sénateurs Fernique monte. Interrogé sur le devoir de vigilance des entreprises.-- Il faut nous féliciter de l'accord que nous auquel nous sommes parvenus jeudi dernier parce qu'il dessine le régime de vigilance le plus ambitieux dans le monde en 2017 et vous l'avez rappelé, la France a été le 1er pays au monde à adopter des règles juridiquement contraignante sur le devoir de vigilance des entreprises et monsieur le président Laurent j'ai je ne partage pas votre pessimisme et d'ailleurs je vous invite à en discuter. Avec Dominique Potier qui avait créé ce groupe transpartisan et avec elle, nous avons beaucoup et avec qui nous avons beaucoup échangé pendant ce processus. La France a très fortement soutenu ce projet de directive européenne. Et fort de son expérience puisque c'est le 1er pays avec un cadre aussi étendue, a plaidé pour un cadre de vigilance ambitieux et opérationnel au niveau européen. Vous l'avez rappelé, messieurs les sénateurs, cette ambition aurait encore pu être plus forte. Sur la santé et la sécurité des travailleurs. Sur les sociétés mères des grands groupes des multinationales, ou encore sur la responsabilité civile des entreprises. Mais l'Union européenne suppose des compromis et nous avons eu toutefois confiant conscience et j'étais à nouveau à ce qu'on que l'équilibre au Conseil ne permettait pas d'atteindre tous ses objectifs et nous espérons que les discussions avec le Parlement européen permettront d'améliorer encore ce texte enfin et je vais pouvoir clarifier ce point, la France n'a jamais demandé l'exclusion des services financiers de ce texte. Nous avons demandé que le secteur financier soit traité comme tous les autres secteurs de l'économie. Un autre sujet ce sont les ministres de la Justice et des affaires intérieures qui se réuniront à Bruxelles et et plusieurs d'entre vous m'ont parlé des migrations. Jeudi prochain, ils auront l'occasion de revenir sur le plan d'action qui a été décidé lors du conseil extraordinaire du mois dernier, pour mieux gérer les routes migratoires dans les Balkans et en Méditerranée. En ce qui concerne les bateaux. Il a été créé un groupe de contact des États qui va inclure les ONG pour éviter de répéter, monsieur le sénateur Cadec effectivement ce que nous avons vu et qui est à déplorer. Il y a quelques semaines. Vous le savez depuis 2 ans, messieurs les sénateurs, Richard. Je crois, vous avez raison, nous avançons sur le pacte Asile et Migration il a d'ailleurs été débloqués sous présidence française, l'Union européenne. Ça faisait 10 ans qu'il était bloqué. Monsieur le sénateur, et nous avançons avec un autre triptyque. Celui de la solidarité entre les pays de l'Union européenne. C'est essentiel pour la liberté de circulation dans l'espace Schengen et cette solidarité, elle va de Pair avec responsabilité mais aussi la France en a fait preuve il y a quelques semaines avec humanité. Lors du prochain un conseil affaires intérieures. Les ministres évoqueront aussi l'élargissement de l'espace Schengen. Que vous avez de nouveau évoqué. Et les nombreuses évaluations qui ont été réalisées démontrent que la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie appliquent correctement ses règles de Schengen. Elles sont prêtes à rejoindre l'espace Schengen en contribuant de manière positive à sa sécurité. Les traités prévoient et vous le savez, que la décision politique de cette pleine intégration appartient désormais au conseil à l'unanimité. Et à l'heure où nous parlons cette unanimité ne semblent pas réunies, la présidence travaille donc pour parvenir à un consensus sur cette question un consensus qui peut aussi être un compromis. Madame la présidente Gruny, vous me pardonnerez de vous ramener le taux aussi ostensiblement et madame la sénatrice. Guillotin, vous m'avez interrogé sur l'Europe de la santé. Je la cherche et de la stratégie pharmaceutique.-- C'est effectivement un enjeu particulièrement important pour la France puisqu'ils participent au renforcement de notre autonomie stratégique européenne. Et la révision de la législation pharmaceutique de l'Union doit être présenté par la Commission en décembre prochain. Nous sommes assez confiants, nous pensons qu'elle répondra à cet enjeu. Concernant l'espace européen de santé donc des entreprises qui pourraient être en charge du stockage des données. Les discussions sont encore en cours. Au Conseil. Le contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont produit un avis sur la question et comme vous le savez sûrement, ils ont noté. Notamment proposé qu'il soit inscrit dans le texte que ces données doivent être hébergés sur le territoire de l'Union européenne.-- Vous l'avez dit, monsieur le sénateur Gattolin mais aussi messieurs les sénateurs Marie-. Jamais l'union n'aura autant avancer que ces derniers mois en matière de robes d'union des marchés de l'énergie de lutte contre les ingérences étrangères et sur l'ensemble de ces sujets, le maître mot je crois et celui de souveraineté. Ce même agenda de souveraineté que le président de la République, il avait proposé à nos partenaires européens dès 2017 dans le discours de la Sorbonne. Ce mot souveraineté, il est aujourd'hui repris, y compris par nos partenaires, de même que celui de boussole ou d'autonomie stratégique. C'est dire. Et je crois qu'il faut vraiment le saluer comme vous l'avez fait ce soir l'ampleur du changement du paradigme qui s'est opéré depuis lors. Alors oui, l'Europe avance d'autant plus vite face aux crises. Et il en est je crois de notre responsabilité commune oui, l'Europe est complexe et l'on n'avance pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait, mais nous sommes 27. Hein. Construire cette Europe. Et vous l'avez souligné madame la sénatrice Jourda. Je crois que c'est l'honneur de la France. Parmi ses 27 que d'être constamment à l'initiative et force de proposition, je vous remercie. Merci madame la ministre. Alors pour conclure le débat. La parole est à monsieur Jean-François Rapin, président de la commission des Affaires européennes pour cinq minutes. Merci madame la présidente, moi aussi je vais vous tournez le dos ostensiblement quelques instants de depuis le bas mais rassurez-vous, seulement quelques instants. Pour conclure cette cette session ma madame la mini-je vous remercie d'avoir répondu aussi précisément et nominativement. À à tous les sénateurs qui qui sont venus ce soir et qui sont intervenus sur des sujets très importants, très intéressant dont on a l'impression finalement qu'ils sont redondants parce que rythmé rythmée par la guerre en Ukraine et ça depuis un certain temps. Mais c'est tellement important et je voudrais juste revenir sur 2 points. Le 1er c'est celui. Qu'on a évoqué au travers la justice qui devra un jour se porter. À l'encontre des des crimes qui sont perpétrés par les Russes. Mais au-delà des crimes physiques tels qu'on les a ressenties telles qu'on les voit tels qu'ils sont. Présentés par les médias. Il y a aussi. Ce Crime majeur qui nous a été exprimée par les députés. Qui sont venus nous voir la semaine dernière. Qui sont ceux de la déportation. Et là je pense que. Aussi bien vice-président Alizard s'est exprimé sur ce qui peut se passer en Birmanie, demain. Moi je dis aussi ce qui peut se passer dans dans les mois et les années à venir avec toutes ces tous ces enfants qui ont été déportés. Toutes ces familles. L'Europe doit avoir un regard très particulier. L'Union européenne doit avoir un revers très très particulier sur cette situation. Pour le moins dramatique.

Je pense et là je le dis en tant que professionnel de santé. J'ai reçu aujourd'hui un nombre d'alertes considérable. À la fois des professionnels, délivrant les médecins sont entre autres les pharmaciens mais aussi des patients qui nous explique. Il est même difficile d'avoir des antibiotiques là en ce moment. Dans les pharmacies, donc il y a il y a vraiment un réel problème, mais c'est un problème récurrent et cyclique, on l'a évoqué ici, moi je me souviens avoir posé, je ne sais 2 ou 3 questions d'actualité sur le sujet. Et pour des produits tout à fait différent. On a eu un problème avec les antihypertenseurs puis après avec les corticoïdes là aujourd'hui ce sont les antibiotiques. Attention à ça. Attention à ça. Ne remettons pas. Une 2ème crise sanitaire sur la crise sanitaire que nous venons de de vivre parce qu'on manquerait de on manquerait de de traitement et de médicaments, on pense toujours que ça arrive aux autres, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui qui pousse, puis un 3ème point évoquiez. J'ai encore un tout petit peu de temps et je ne vais pas l'utiliser. C'est la question de la la communauté politique européenne. Sincèrement au tout début je pensais que ça pouvait être un outil gadgets. Ben on se rend compte au fil des rencontres qu'on peut avoir avec. Nos collègues qui qui l'intègre progressivement. Que ça peut être ou quelqu'un outil intéressant mais je pense que le message à faire passer à toutes ces nations qui veulent entrer dans cette communauté politique européenne, que c'est à elle de le la faire vivre aussi. Elles ne peuvent pas attendre tout de l'Union européenne elle ne peuvent pas attendre tout des États membres et elles doivent pouvoir aussi émerger et faire leurs propres propositions, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs j'étais en déplacement avec le président l'archi en Serbie. Récemment, et voilà donc on la CPE n'est n'est pas. Un nouveau paradis aussi ça doit être un outil. Voilà donc je pense qu'on peut. Conclure là-dessus, on vous remercie encore Madame la Ministre. Bonne soirée à tous. Merci monsieur le président. Nous en avons terminé avec ce débat. Mais, chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance mercredi 7 décembre à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. Et la séance est levée.